nos anciens collègues André Dulait, qui fut sénateur des Deux-Sèvres de 1995 à 2014 et qui fut aussi président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, et des forces armées, et Bernard Joly, qui fut sénateur de la Haute-Saône de 1995 à 2004.

la séquence qui s'ouvre aujourd'hui revêt une dimension singulière par les thèmes que nous allons aborder. Chacun mesure l'importance des échanges que nous allons avoir, et c'est avec beaucoup d'humilité que nous entamons l'examen de ce texte. Ne nous y trompons pas, les projets de loi relatifs à la bioéthique, s'ils peuvent sembler techniques, voire abstraits, recouvrent des enjeux très concrets qui touchent au plus profond de l'intimité des Français la famille, l'enfance, la maladie et tout ce qui compose une vie dans ses choix ou dans ses espoirs. C'est donc à une réflexion profonde que vous êtes invités, que nous sommes invités. Une réflexion non pas sur des problèmes à résoudre ou sur des défis à relever, mais bien sur la société dans laquelle nous voulons vivre et la société que nous voulons proposer aux générations futures. La France prend rendez-vous à intervalles réguliers avec les grandes questions de notre temps, avec le champ des possibles ouvert par la science et la recherche biomédicale. Ce champ des possibles est vaste, mais nos principes sont solides. Ces principes sont autant de jalons et de limites à ne pas dépasser. Ces grands principes, ils sont au coeur du projet de loi : la dignité de la personne humaine, l'autonomie de chacun et la solidarité de tous. Ces grands principes ne sont pas des verrous, ce sont des balises qui nous guident et nous protègent. Nos choix refléteront nécessairement un certain état de la science, de la société, des mentalités et, évidemment, de l'éthique. Ces choix sont ceux de la confrontation entre le possible et le souhaitable, entre des parcours individuels, parfois douloureux, et des conséquences collectives acceptables. Ces choix, nous les ferons ensemble, parce que c'est au Parlement, et nulle part ailleurs, qu'ils doivent être faits.

Le Prométhée définitivement déchaîné, auquel la science confère des forces jamais encore connues et l'économie son impulsion effrénée, réclame une éthique qui, par des entraves librement consenties, empêche le pouvoir de l'homme de devenir une malédiction pour lui. » Nous ne sommes pas réunis pour autre chose. Les thèmes qui vont nous mobiliser sont exigeants, passionnants et s'accommodent mal des raccourcis et des caricatures. Le projet de loi que je vous présente aux côtés de Nicole Belloubet, de Frédérique Vidal et d'Adrien Taquet a été largement nourri par vos travaux parlementaires. Il a aussi été enrichi à l'Assemblée nationale et par les travaux de la commission spéciale de votre assemblée. Il le sera encore par les débats qui s'ouvrent aujourd'hui. Ce long cheminement n'a rien d'anodin ; il était et reste nécessaire. La méthode retenue depuis plusieurs mois a été, je crois, à la hauteur de l'enjeu, c'est-à-dire à la hauteur de ce que nous sommes, ni plus ni moins des hommes et des femmes avec leur histoire personnelle, leur sensibilité et leur sens du bien commun devant des choix qui vont structurer la société française de demain. C'est dans ce même esprit que nous allons avancer dès aujourd'hui pour adapter notre droit, non pas à une société post-moderne tantôt espérée, tantôt redoutée et souvent fantasmée, mais à la société telle qu'elle est ici et maintenant, et surtout aux Français tels qu'ils sont ici et maintenant, dans leur très grande diversité. Accéder à des techniques médicales et accorder de nouveaux droits, ce n'est pas déréguler ; c'est au contraire permettre à la République de tenir compte des avancées scientifiques et médicales et de s'adapter à la vie des Français. J'aurai l'occasion de revenir devant vous à plusieurs reprises pour présenter certaines dispositions et débattre ensemble de leur contenu. Le projet de loi travaillé par la commission spéciale porte toujours les avancées que le Gouvernement a proposées en matière de procréation d'une part, l'ouverture de l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées ; d'autre part, l'autorisation de l'autoconservation des gamètes. Ces mesures majeures ont été approuvées par les sénateurs et je m'en réjouis. Ces nouvelles dispositions doivent néanmoins être parfaitement encadrées et nous y veillerons avec la plus grande rigueur. Ces mesures ouvrent des droits. Ces droits sont effectifs chez la plupart de nos voisins européens ; ils ne sont contraires à aucun principe de la bioéthique et ils peuvent être exercés dans un cadre protecteur, en particulier pour l'enfant à naître. L'ouverture de ces droits, c'est l'ouverture sur un avenir que nous regardons avec confiance. Soyons lucides : les familles monoparentales et homoparentales existent déjà elles sont issues de projets souvent très longs avec des enfants qui sont ardemment désirés et des parents, nul ne s'en étonnera, qui sont des parents, tout simplement. Je veux couper court à une idée fausse : il n'y a pas, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de droit à l'enfant. Tout projet parental formulé dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation est déjà, dans le droit en vigueur, soumis au respect de l'intérêt de l'enfant à naître ; et il continuera de l'être. Reconnaître la famille dans ce qu'elle a de divers, de pluriel et de riche, c'est ce que nous vous proposons.

Nous savons que l'anonymat du donneur a bien souvent pour corollaire le silence des parents et des questions sans réponse de l'enfant. Permettre à l'enfant d'accéder à sa majorité à des informations relatives au donneur, c'est lui permettre de se construire comme individu, de se pacifier avec son histoire et, donc, avec lui-même. Un donneur n'est pas un parent, ce n'est pas sa vocation, ce n'est pas le sens de son geste. Mais il est une pièce de son identité que l'on ne peut dérober à l'enfant, il est un chaînon qui ne doit pas manquer à l'appel d'une existence. Donner accès aux origines par ce projet de loi, c'est aussi sortir le don du secret pour le reconnaître dans ce qu'il a de profondément humain, altruiste et solidaire. Ce faisant, nous n'affirmons qu'une seule chose : la force des institutions qui encadrent et qui protègent chacun. Nous ne ferons qu'un seul choix, celui de la responsabilité individuelle et collective. Le projet que nous examinons comprend aussi de nouvelles mesures en matière de génétique auxquelles je suis fondamentalement opposée. Le séquençage à haut et très haut débit de l'ADN a révolutionné le domaine de la génétique. Le projet de loi initial proposait des mesures concrètes pour accompagner l'augmentation des indications et des usages des examens génétiques réalisés dans le cadre du soin ou dans le cadre de la recherche. Mais la facilité et la rapidité d'analyse du génome permettent aisément de dépasser ce cadre. Toutes les mesures dont nous allons parler- dépistage génétique en population générale, dépistage préconceptionnel, dépistage préimplantatoire, dépistage génétique néonatal -sont en effet intimement liées. Ces mesures peuvent paraître positives ; mais, derrière elles, que cherchons-nous à prévenir ? Le dépistage en population vise à connaître les maladies auxquelles on serait prédisposé. Que fait-on de l'absence de preuve de l'utilité médicale d'une telle démarche ? Que fera-t-on de ces résultats que l'on ne sait pas interpréter et qui amèneront la personne à se méprendre sur son état de santé, présent comme futur ? Le dépistage préconceptionnel ouvert à tout couple en âge de procréer vise à identifier le risque d'avoir un enfant atteint de certaines maladies. Mais comment définirons-nous ces maladies ? Au regard de la mortalité ? Au regard du handicap ? Par ailleurs, l'expression d'une mutation est variable et l'on ne sait pas le prédire à ce jour. Il s'agit donc d'éviter la naissance d'enfants sur la base d'une anomalie génétique dont on ne peut prédire comment elle s'exprimera. Que penser de notre modèle de société inclusive si l'on ne veut plus prendre le risque de la différence ? Quel impact sur les couples qui feront les tests ou, au contraire, qui ne les feront pas ? Quel impact sur la diversité génétique de notre espèce ? On peut tirer le fil pour toutes ces mesures. Mais une chose est certaine : le généticien ne doit pas se substituer à la Pythie grecque que l'on interrogeait pour connaître son avenir ; des examens médicaux ne sauraient devenir des oracles parce que la vie n'est jamais réductible à une prédiction, aussi scientifique soit-elle. C'est pourquoi nous sommes convaincus que le temps est à la recherche pour mieux comprendre l'impact des différentes mutations et leurs conséquences en termes de prévention, de soins et de société. Dans le champ du dépistage préimplantatoire des aneuploïdies, qui sont une anomalie du nombre de chromosomes, comme les trisomies, l'objectif peut paraître louable il est d'améliorer l'efficacité des fécondations en évitant le transfert des embryons non viables, et donc capables de générer des fausses couches. Mais, sur le plan scientifique et médical, l'efficacité de la technique est discutée et il est indispensable de poursuivre les recherches avant de modifier la loi. D'ailleurs, un projet de recherche a été sélectionné et sera financé, dès 2020, dans le cadre du programme hospitalier de recherche clinique. Au-delà de l'objectif d'amélioration de la procréation médicalement assistée, il ne faut pas occulter le débat : l'enjeu, une fois la technique autorisée, sera également la réimplantation ou non d'embryons viables, mais présentant des anomalies génétiques. Pour moi, les risques sont réels et les bénéfices incertains. Si nous soutenons l'effort et l'essor de la médecine génomique dans un cadre médical et sécurisé, le Gouvernement n'est pas favorable à une libéralisation de l'accès aux tests génétiques. je vous alerte, enfin, sur les tests généalogiques dits « récréatifs ». Les tests généalogiques exposent à une multitude de risques peu connus, mais qui constituent une menace sérieuse pour la vie privée des consommateurs. Si l'objectif est de rechercher d'éventuelles proximités de parenté, cela a un impact sur d'autres membres de la famille, qui n'y ont donc pas consenti. La démarche des sociétés qui proposent ces tests n'est pas philanthropique : elle est d'abord commerciale, et la généalogie est le plus souvent un cheval de Troie qui ouvre la voie au dépistage génétique à visée médicale dont je parlais à l'instant. Face à vous, je serai déterminée. Ces sujets ne laissent pas indifférents, ces sujets nous obligent à un débat parlementaire exigeant, serein et apaisé. Nous avons fait le choix, non d'engager la procédure accélérée, mais bien de laisser à chacun, dans chacune des chambres, le temps de débattre et de modifier le texte. De la même manière, le Gouvernement prend acte des modifications qui sont intervenues en commission spéciale. Certaines posent des questions techniques, d'autres plus politiques. Nous avons souhaité déposer des amendements sur les seuls éléments que nous considérons comme des lignes rouges à ne pas franchir pour garantir l'équilibre du projet de loi. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, un grand projet collectif nous attend : le projet d'une société en phase avec elle-même, d'une société qui reconnaît des droits nouveaux, sans rien céder aux principes qui nous lient les uns aux autres. Dans les prochaines semaines, vous serez des artisans et des garants : les artisans d'un droit qui s'adapte à la France et aux Français du XIX siècle, les garants d'un projet qui protège et qui émancipe. C'est ce projet collectif qui nous réunit aujourd'hui. La parole Monsieur le président, monsieur le président de la commission spéciale, mesdames, messieurs les rapporteurs, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, j'ai le plaisir, aux côtés d'Agnès Buzyn, de Frédérique Vidal et d'Adrien Taquet, de vous présenter aujourd'hui ce texte important de révision des lois bioéthiques. En tant que membre du Gouvernement, je suis bien entendu particulièrement fière de co-porter cette loi, qui, dans son ensemble- Agnès Buzyn vient de le rappeler -, réaffirme des principes et des valeurs, mais traduit aussi de véritables progrès. Je pense notamment à son article 1, qui ouvre l'assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes seules. Je me réjouis donc que la commission spéciale ait décidé de repousser les amendements de suppression de l'article 1 du projet de loi. Je souhaite évidemment qu'il puisse en être de même en séance publique. Cela répond en effet à une réalité sociologique qui ne peut être ignorée ; elle est liée à la pluralité des situations familiales. En tant que garde des sceaux, je suis plus particulièrement chargée de l'article 4 de ce projet de loi, qui tire précisément les conséquences, sur le plan de la filiation, de l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes. Cette question de l'établissement de la filiation des enfants nés au sein de couples de femmes ayant recours à une PMA avec tiers donneur suscite à la fois des interrogations et des débats légitimes. Plusieurs options étaient envisageables sur ce point. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Gouvernement avait saisi le Conseil d'État. Je rappelle brièvement quelles sont les options qui pouvaient être offertes d'une part, une extension des dispositions de droit commun, même si ces termes de droit commun sont impropres ; d'autre part, la création d'un dispositif applicable à l'ensemble des couples, hétérosexuels comme homosexuels, qui avaient recours à une PMA avec tiers donneur ; ou encore la création d'un dispositif applicable aux seuls couples de femmes ayant recours à la PMA avec tiers donneur. de ces options, présente des avantages et des inconvénients qui vous ont très certainement été largement exposés dans le cadre des auditions que vous avez menées. Ce qui a présidé au choix du Gouvernement, ce sont les quatre principes et objectifs suivants. Il s'agissait d'abord pour nous d'offrir aux enfants nés d'AMP au sein d'un couple de femmes les mêmes droits que ceux qui sont offerts aux autres enfants. C'est un choix d'égalité qui est évident, mais qui devait être ici affirmé et réaffirmé fortement. Deuxième objectif : apporter la sécurité juridique aux deux mères et à leurs enfants. La filiation, dans cette hypothèse précise, peut être établie non sur la vraisemblance biologique, mais sur la base d'un engagement commun. C'est donc une évolution juste, mais elle doit être juridiquement solide. Troisième objectif il s'agissait pour nous de construire une procédure simple, qui n'impose aucune démarche supplémentaire pour les couples de femmes pour l'établissement de leur filiation. Enfin, quatrième objectif : il s'agissait de ne pas revenir sur le droit applicable aux couples hétérosexuels. Nous souhaitons en effet ouvrir des droits nouveaux sans rien retirer ou modifier du régime de filiation applicable aux couples hétérosexuels. C'est donc sur la base de ces quatre principes clairs que nous avons fait le choix d'un dispositif pour l'établissement de la filiation pour les couples de femmes ayant recours à l'AMP avec tiers donneur. Le dispositif proposé par le Gouvernement dans le projet de loi initial a été enrichi dans le cadre des débats à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, de manière très concrète, il se présente de la façon suivante. D'abord, les couples de femmes doivent consentir devant notaire à faire une PMA avec tiers donneur, comme c'est aujourd'hui le cas pour les couples hétérosexuels. Au même moment, lors de ce même entretien devant le notaire, elles s'engagent à devenir les mères de l'enfant qui naîtra. Cette reconnaissance conjointe sera produite lors de la naissance devant l'officier d'état civil en même temps que le certificat d'accouchement, ce qui permettra d'établir la filiation à l'égard des deux mères. L'acte intégral de naissance de l'enfant comportera la mention qu'il a été reconnu conjointement par les deux mères. Ce dispositif a évolué au cours du travail mené avec les rapporteurs à l'Assemblée nationale. Les modifications, qui ne remettent pas en cause les objectifs que j'ai rappelés plus haut, ont porté essentiellement sur deux points.

avait créé un nouveau titre VII propre à la filiation des enfants nés de couples de femmes ayant recours à l'AMP, le dispositif finalement adopté à l'Assemblée nationale est intégré au sein du titre VII du livre I du code civil relatif à la filiation.

Ce chapitre nouveau est toutefois très précisément organisé. Il comporte d'abord les dispositions communes- interdiction d'établir un lien de filiation avec le donneur, condition et forme du consentement -, puis les dispositions qui permettent l'établissement de la filiation dans les couples de femmes. Ce déplacement par rapport au projet initial du Gouvernement permet de rendre compte du socle commun entre ces modes de filiation. Il permet donc de rapprocher autant qu'il est possible les modes d'établissement de la filiation des couples de femmes et des couples hétérosexuels qui ont recours à l'AMP avec tiers donneur. Pour autant, ce nouvel emplacement ne bouleverse pas le droit de la filiation dès lors que les quatre premiers chapitres du titre consacrés à la filiation reposant sur la vraisemblance biologique, ne sont pas modifiés. Je le répète : les couples hétérosexuels ayant recours à l'AMP avec tiers donneur ne voient pas modifié l'établissement de leur filiation. La seconde évolution qui a résulté des débats conduits à l'Assemblée nationale concerne la notion de reconnaissance conjointe. Dans le projet de loi initial, le Gouvernement avait proposé d'établir une déclaration anticipée de volonté (DAV).

juridique, voire un objet juridique nouveau, qui, aux yeux de certains, pouvait être considérée comme stigmatisante pour les couples de femmes. Là encore, et cela a son importance, le Gouvernement assume au maximum la volonté de réduire la différence entre les couples hétérosexuels et les couples de femmes, tout en respectant l'exigence de sécurité juridique. Il n'y a en effet aucune confusion possible entre cette reconnaissance conjointe et la reconnaissance de l'article 316 du code civil la première est donc conjointe, effectuée avant même la grossesse, tandis que la seconde est unilatérale et effectuée après la naissance ou, au plus tôt, au début de la grossesse. La reconnaissance conjointe n'est possible que pour les couples de femmes, tandis que la reconnaissance de l'article 316 n'est pas ouverte aux couples de même sexe. Pour établir une double filiation maternelle, l'officier d'état civil devra donc exiger cette reconnaissance conjointe, ainsi que le certificat d'accouchement. Il n'y a dès lors aucune confusion possible entre ces deux modes d'établissement de la filiation. Concrètement, je l'ai déjà dit, l'acte de naissance de l'enfant portera la mention qu'il a été reconnu conjointement par les deux mères. Cette mention attestera bien que l'on est dans l'hypothèse légale d'une double filiation maternelle. Ainsi, grâce à son double caractère- elle est simultanée et anticipée -, cette reconnaissance conjointe permet de sécuriser la filiation, particulièrement à l'égard de la femme qui n'accouche pas. Les deux femmes seront mères en même temps, à égalité, dès lors que l'accouchement aura eu lieu. La reconnaissance conjointe permet donc de faire obstacle à l'éventuelle reconnaissance par un tiers avant la naissance, puisque cette reconnaissance conjointe lui sera en tout état de cause antérieure et qu'elle primera devant l'officier d'état civil. Ce dispositif simple est donc particulièrement sécurisant, pour les enfants comme pour les mères- c'était la première de nos exigences. À la faveur des débats, un autre sujet s'est imposé à nous au cours de la navette parlementaire : la gestation

liminaire. D'abord, l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules ne peut ni ne doit en aucun cas conduire à autoriser la GPA au nom du principe de non-discrimination. En effet, le principe d'égalité ne trouve pas, en l'occurrence, à s'appliquer. D'abord, parce qu'il n'existe pas de droit à l'enfant. ! D'autre part, parce que, au regard de la procréation, les couples de femmes et les couples d'hommes ne sont pas dans une situation identique. Ensuite, la reconnaissance la reconnaissance du désir d'enfant pour les couples d'hommes ou les hommes célibataires soulève des enjeux totalement différents de ceux qui sont liés au recours à la PMA. Pour la GPA, le degré d'implication du tiers, sans commune mesure avec celui du donneur de gamètes, est tel qu'il porte atteinte aux principes, que nous avons maintes fois réaffirmés, de non-marchandisation du corps humain et d'indisponibilité de l'état des personnes.

lorsque des couples se rendent à l'étranger pour recourir à une GPA et qu'ils rentrent en France avec les enfants nés de cette gestation pour autrui, l'État doit garantir à ces enfants une vie familiale normale, ainsi qu'une filiation reconnue dans notre état civil. Je prête donc une attention toute particulière à la question de l'établissement du lien de filiation des enfants nés de GPA à l'étranger. Dans ses arrêts récents, du 18 décembre dernier, portant sur la transcription des actes d'état civil étrangers établis à la suite d'une GPA réalisée à l'étranger, la Cour de cassation

juge, désormais, que la conformité à la réalité d'un acte d'état civil étranger s'apprécie au regard des critères de la loi nationale étrangère, non de ceux de la loi française. Cette solution est source de difficultés, car elle soustrait les GPA réalisées à l'étranger au contrôle du juge français, s'agissant en particulier de l'intérêt de l'enfant et de l'absence de trafic d'enfants. De fait, il n'est plus nécessaire de prévoir une adoption pour reconnaître le lien de filiation.

Dans ce domaine, il faut exclure toute généralisation dont la portée n'aurait pas été mesurée avec soin. Il faut savoir protéger les enfants

sécurisant, réaliste et juridiquement solide, qui offre à tous les enfants les mêmes droits et à leurs parents les mêmes droits et les mêmes devoirs, quelle que soit leur orientation sexuelle. En toute hypothèse, je serai extrêmement attentive à nos débats et à nos échanges. La parole

Monsieur le président, monsieur le président de la commission spéciale, mesdames, messieurs les rapporteurs, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, le débat qui s'ouvre

la bioéthique- cela a été dit -n'est pas une affaire de spécialistes, juristes ou scientifiques : c'est une série d'enjeux et d'interrogations, un questionnement, que nous avons tous en partage. Avoir institué le réexamen périodique de la loi de bioéthique est une spécificité nationale tout à fait remarquable. Chacune des lois intervenues depuis 1994 a permis de faire se rencontrer la société et les avancées de la science.

exigence. Notre discussion se fonde sur un principe auquel nous souscrivons tous : ce que la science sait rendre possible n'est pas nécessairement aligné sur le souhaitable. Pourtant, chacun mesure au quotidien à quel point les progrès scientifiques réalisés ces dernières années interrogent nos cadres habituels de pensée, qu'il s'agisse de la recherche sur l'embryon, sur les cellules souches embryonnaires ou induites, ou en matière génétique. Combler ce hiatus et résoudre cette tension entre les propositions de la recherche et les aspirations de notre société, c'est le coeur même de notre droit de la bioéthique. Le Sénat joue un rôle considérable, depuis 1994, dans la construction de ce droit, et je ne crois pas me tromper en affirmant que l'ensemble de la communauté de la recherche sait ce qu'elle doit à la Haute Assemblée, s'agissant de l'instauration, en 2013, du régime d'autorisation en matière de recherche sur les cellules souches embryonnaires. Je l'ai déjà rappelé devant la commission spéciale, mais il me semblait important d'y insister aussi à cette L'encadrement de la recherche est un travail de funambule : il s'agit de ne sacrifier ni nos valeurs fondamentales à une quête éperdue de savoir, ni l'espoir de développer des thérapies innovantes et de guérir des maladies aujourd'hui incurables à des préjugés qui ne correspondent plus à l'état des connaissances. Ainsi, des questionnements initiaux relatifs à la recherche sur l'embryon demeurent, mais actualisés par les percées scientifiques les plus récentes,

repose également sur la manière différente dont les progrès scientifiques les plus récents nous permettent désormais d'interroger le sujet de la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, qui sont au coeur de notre droit de la bioéthique. En matière de recherche sur l'embryon, le projet de loi autorise les chercheurs à conduire des recherches incluant l'édition du génome d'embryons ne faisant plus l'objet d'un projet parental et susceptibles de contribuer au progrès de la connaissance, avant d'être détruits. Ces recherches apportent des connaissances essentielles à la compréhension du rôle de nos gènes dans les mécanismes de différenciation cellulaire à l'oeuvre au cours du développement, mais aussi dans d'autres processus physiologiques ou pathologiques. Auparavant, nous ne savions pas observer ces embryons sur une période supérieure à quelques jours. Les techniques ayant évolué, nous savons désormais les observer à des phases ultérieures de leur développement.

n'est pas arbitraire, ni attachée aux limites de ce que nous savons faire : elle est fondée sur un consensus scientifique international. Le présent projet de loi est donc non pas un blanc-seing donné aux scientifiques, mais la recherche d'un point d'équilibre.

la création d'embryons à des fins de recherche est interdite, de même que la modification du patrimoine génétique transmissible à la descendance ; l'intégration de cellules animales dans un embryon humain est encore plus clairement prohibée.

tout en faisant barrage à toute possibilité de clonage ; il en va de même s'agissant de la modification du patrimoine génétique d'un embryon destiné à être implanté. Toutefois, le projet de loi réserve des espaces propices aux innovations thérapeutiques que nous pourrions mettre au point, si nous comprenions mieux les mécanismes du développement et de la différenciation cellulaire. Ces mécanismes sont au coeur de nombreuses pathologies que nous comprenons parfois mal, faute de concepts scientifiques pour les traiter ; c'est le cas, notamment, des cancers pédiatriques les plus difficiles à traiter, issus de dysfonctionnements dans la différenciation cellulaire-

S'agissant des cellules souches embryonnaires, leur capacité à se transformer en n'importe quel type de cellules du corps humain ouvre de grandes perspectives à la thérapie cellulaire et à la médecine régénérative.

diabète. Seulement, le régime juridique auquel la recherche sur ces cellules est actuellement soumise pèse considérablement sur l'avancée des travaux des chercheurs, car il se confond avec celui qui encadre la recherche sur l'embryon, alors même qu'embryon et cellules souches embryonnaires ne relèvent plus du même questionnement éthique. En effet, nous maîtrisons aujourd'hui les techniques avancées permettant de dériver des lignées, très longues et parfois très anciennes, de cellules souches. Celles qui sont étudiées aujourd'hui dans les laboratoires français sont majoritairement issues de lignées dérivées voilà plus de vingt ne résultent donc pas d'un nouvel embryon. De ce fait, ce qui interpelle aujourd'hui est moins l'origine des cellules souches que notre capacité à dériver les lignées actuelles sans les altérer et en conservant leur potentiel pluripotent. Notre capacité à dériver ces cellules souches n'épuise naturellement pas la nécessité de poursuivre la recherche sur l'embryon : il va de soi que nos chercheurs auront besoin de produire de nouvelles lignées de cellules souches. À cet égard, je tiens à rassurer la Haute Assemblée sur l'un des nombreux principes qui encadrent notre recherche : jamais un embryon n'est créé à des fins de recherche- il faut être très clair sur ce sujet. Nombreux sont ceux qui craignent qu'on emploie les cellules souches pour produire des gamètes et, partant, des embryons artificiels. Les embryons destinés à la recherche sont issus de dons, à la suite d'un projet parental : ce principe fondateur n'a pas vocation à être remis en cause. À ce jour, un peu moins de 3 000 embryons ont été proposés et utilisés à des fins de recherche depuis 1994, tandis que près de 19 000 ont d'ores et déjà fait l'objet d'un don à la science.

Le présent projet de loi rend également compte de la manière dont le législateur peut se saisir de l'actualité scientifique la plus récente, au travers de la question des cellules souches pluripotentes induites.

Il s'agit de cellules adultes que nous savons faire évoluer jusqu'à un stade très proche de celui des cellules souches embryonnaires. Je dis : très proche, car si les cellules souches embryonnaires disposent de la capacité à produire tout autre type de cellules de l'organisme, les cellules souches pluripotentes induites ont un caractère pluripotent plus limité. si les cellules souches embryonnaires peuvent devenir n'importe quelle autre cellule humaine, ce n'est pas le cas des cellules souches induites, dont les évolutions sont plus limitées, en l'état actuel de la connaissance. Je tiens donc à être très claire aussi sur ce point : si la découverte des cellules souches pluripotentes induites a été un événement scientifique majeur, ces dernières ne peuvent offrir une alternative ni à la recherche sur les cellules souches embryonnaires ni à la recherche sur l'embryon. d'un nouveau territoire de la connaissance que nous vous proposons de faire adhérer au cadre rénové dont le présent projet de loi est porteur, afin que l'Agence de la biomédecine exerce la totalité de ses prérogatives auprès de la communauté scientifique. Qu'il s'agisse de cellules souches embryonnaires ou de cellules souches pluripotentes induites, les travaux de la commission spéciale ont mis en exergue la problématique des embryons chimériques, sur laquelle il me paraît fondamental de revenir quelques instants.

discussion. Les chimères ne résultent pas de manipulations génétiques : il s'agit non pas de modifier le génome, mais d'observer les évolutions cellulaires d'un embryon animal auquel sont agglomérées des cellules souches embryonnaires ou induites. question non pas de franchir la barrière des espèces, ... Alors, c'est quoi ? ... mais d'observer, dans des cadres différents, les mécanismes de différenciation qui sont au coeur de la recherche sur l'embryon et les différentes catégories de cellules souches. Le cadre législatif actuel en matière de bioéthique interdit l'introduction de matériel génétique animal dans un embryon humain : cette interdiction absolue est bien rappelée dans le texte qui vous est soumis.

à des techniques sur lesquelles de grands espoirs sont fondés. Au-delà de l'imaginaire charrié par la notion de chimère, ce qui est en jeu, c'est bien notre capacité à continuer à disposer de modèles animaux nous permettant de mieux comprendre certaines pathologies humaines et leur traitement ; c'est de cela qu'il s'agit, ni plus ni moins. Beaucoup a été écrit sur certains protocoles de recherche annoncés au Japon. Ce qui est scientifiquement établi, c'est que, à ce jour, nos connaissances ne nous permettent pas de conduire ces embryons jusqu'à la parturition ; il est tout aussi établi que nous ne savons pas utiliser des embryons animaux pour produire des organes compatibles avec l'homme, ce qui poserait du reste d'importantes questions, éthiques bien sûr, mais aussi sanitaires. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, et ce n'est pas ce qui est en jeu dans le présent projet de loi. de loi. Ainsi, c'est en ouvrant de nouvelles voies et en traçant de nouvelles limites, en réaffirmant des lignes rouges, que ce texte dessine les contours d'une recherche libre et responsable.

questions. Le Gouvernement entend que le débat se poursuive dans les conditions de sérénité nécessaires pour que nous puissions, avec l'Assemblée nationale, parvenir à un équilibre sur ces différentes questions.

ceux qui constituent des lignes rouges, du moins des points susceptibles de déséquilibrer le texte ou de l'entraîner dans une direction qui ne nous semble pas opportune, s'agissant notamment du délai d'observation des embryons, du cadre législatif relatif aux chimères

Monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues, accueillir les innovations médicales au service de nos concitoyens et dans le respect des principes éthiques : tel est l'équilibre recherché par la commission spéciale en matière de recherche et de génétique. Dans ce domaine, le texte du Gouvernement nous a semblé ambigu : d'un côté, il ouvre la voie à des expérimentations discutables sur le plan éthique, comme les embryons transgéniques ou chimériques ; de l'autre, il reste en retrait de certaines recommandations du CCNE (Comité consultatif S'agissant de la recherche, la principale novation réside dans un assouplissement du régime des recherches sur lescellules souches embryonnaires : il est pris acte que, n'étant pas des embryons, elles ne doivent pas être soumises aux mêmes règles. En revanche, le projet de loi ne sécurise en rien les recherches sur l'embryon, que les lois de bioéthique ont clairement autorisées mais qui continuent de faire l'objet de contentieux systématiques. Devant ce constat, la commission spéciale a choisi de préciser les prérequis applicables à ces recherches, qui s'inscrivent généralement dans une démarche de recherche fondamentale, dont, par définition, les résultats et les possibles applications cliniques ne peuvent être anticipés. La commission spéciale a également souhaité que la recherche française puisse prétendre à l'excellence dans la compréhension des mécanismes du développement embryonnaire. C'est pourquoi elle a étendu à vingt et un jours la durée limite de développement d'embryons surnuméraires, sur dérogation accordée par l'Agence de la biomédecine. la limite de quatorze jours est aujourd'hui réinterrogée, pour permettre des recherches indispensables à une meilleure connaissance du processus de différenciation des cellules souches embryonnaires. De façon assez surprenante, le texte issu de l'Assemblée nationale normalise des recherches qui soulèvent pourtant des questions éthiques majeures, s'agissant en particulier de la création d'embryons chimériques.

transgression d'une ligne rouge dans le franchissement de la barrière des espèces. Très bien ! Dans ces conditions, la commission spéciale a rétabli l'interdiction de constitution d'embryons chimériques impliquant l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines. Consciente de ce que permet le droit en vigueur, elle a également posé des verrous aux expérimentations impliquant l'insertion de cellules souches pluripotentes humaines induites dans un embryon animal. Même les États-Unis, dont la tradition d'éthique biomédicale est différente, interdisent la poursuite à terme de la gestation d'embryons chimériques ; je ne vois donc pas pourquoi nous autoriserions une telle perspective dans notre pays. sur le sujet sensible du diagnostic préimplantatoire, la commission spéciale a élargi, à titre expérimental, les indications médicales de recours à cette technique, dans le seul objectif d'améliorer la prise en charge de femmes en assistance médicale à la procréation, en évitant des échecs répétés et douloureux.

des questions se posent- j'en aborderai, rapidement, trois. En tout cas, il en est une qui, je crois, ne se pose pas : celle de la légitimité de la demande des femmes qui veulent recourir à l'assistance médicale à la procréation. Le désir d'une femme d'avoir un enfant, quelle que soit sa situation conjugale, quelle que soit son orientation sexuelle, est parfaitement respectable. De la même façon, il me semble que les capacités d'amour, d'attention, d'éducation d'une femme ne dépendent en aucun cas de sa situation conjugale, ni de son orientation sexuelle.

faut répondre d'abord à quelques questions. La première est celle du rôle que nous voulons voir la médecine jouer. La bioéthique a pour effet- à vrai dire, pour fonction -de fixer des limites à ce que nous pouvons demander à la science. Lorsque nous affirmons que la médecine est là pour combler nos désirs, ne renonçons-nous pas au rôle même de la bioéthique, puisque le désir est sans limite ? La deuxième question posée, importante, a trait au sort que nous faisons aux enfants que, dans le cadre de cette extension de l'assistance médicale à la procréation, nous faisons naître

ne disposons- j'en suis navrée -d'aucune étude scientifique véritablement fiable. Certes, un certain nombre d'études sont visées dans l'étude d'impact du Gouvernement,

la naissance. Enfin, la troisième question que nous pouvons nous poser- et qui peut paraître plus technique -concerne le droit de la filiation. Ce dernier est un droit d'ordre public, car c'est celui qui structure la société. Il n'est pas confié aux citoyens : il est réglé par l'État.

Or la volonté est infinie, mais elle est aussi fragile. Devons-nous structurer la société sur un fondement aussi fragile que celui de la volonté ? Voilà, me semble-t-il, les questions que nous devons nous poser et auxquelles nous devons répondre. Le désir d'enfant est respectable, mais la médecine a-t-elle pour rôle de satisfaire nos désirs ? Suffit-il à un enfant d'être l'objet de l'amour et du désir ? Enfin, pouvons-nous structurer la société sur le désir et la volonté ? Voilà ce dont nous serons, entre autres choses, amenés à parler pendant ces débats ! La parole

Comme l'esprit peut hésiter dès qu'il se préoccupe de considérations morales ou éthiques ! » Cette citation, je la fais mienne, car c'est ce que j'ai ressenti tout au long

pour ce qui concerne un certain nombre de dispositions, n'a pas toujours adapté le droit à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques en matière de génétique. Évidemment, ne nous leurrons pas : l'interdiction des tests génétiques en accès libre sur internet est aujourd'hui purement virtuelle. Plus d'un million de Français ont déjà eu recours à ces tests sans avoir aucune garantie que leurs droits étaient protégés. Voilà la réalité ! Leurs données sont librement conservées et utilisées par des sociétés commerciales, qui en tirent profit en monnayant leurs bases de données auprès de laboratoires pharmaceutiques. Des informations médicales sont communiquées sans aucun accompagnement professionnel digne de ce nom, alors même que les personnes recourant aux tests génétiques sur internet le font essentiellement à des fins généalogiques. Interdire par principe sans savoir véritablement interdire a-t-il du sens ? Ne vaut-il mieux pas encadrer ? N'est-ce pas cela la bioéthique à la française : encadrer et humaniser plutôt qu'interdire ? La commission spéciale a pris ses responsabilités. Elle a posé les bases d'un encadrement strict des examens génétiques à visée généalogique, en interdisant la transmission d'informations médicales et en introduisant des garde-fous dans le traitement de données aussi sensibles que les informations génétiques. Suivant les recommandations du CCNE, elle a aussi ouvert la voie à un accès aux examens génétiques en population générale et dans le cadre du dépistage préconceptionnel. Le Gouvernement gardera la possibilité d'établir une liste d'anomalies génétiques « actionnables » pour lesquelles des mesures de prévention ou de soins sont envisageables. S'agissant des embryons chimériques, je partage l'analyse de ma collègue Corinne Imbert. Il convient de poser des limites claires à ce type d'expérimentation pour prévenir tout risque de franchissement de la barrière des espèces, tout en préservant l'excellence de nos équipes de recherche. Enfin, concernant le développement de l'intelligence artificielle, qui constitue également un sujet de première importance, le projet de loi crée opportunément un cadre juridique pour l'utilisation d'un traitement algorithmique lors de la réalisation d'un acte médical. La commission spéciale a renforcé les garanties applicables à l'utilisation de ces technologies, en prévoyant que le patient soit informé en amont de l'utilisation d'un traitement algorithmique et qu'aucune décision médicale ne puisse exclusivement se fonder sur un tel traitement. Mes chers collègues,

Cet aménagement du don du vivant n'a connu qu'une mise en oeuvre timide depuis la précédente loi de 2011. Pour atteindre les objectifs ambitieux du plan Greffe, alors que cinq cents personnes meurent chaque année dans notre pays faute de greffe d'organes, les défis sont encore devant nous. Face à ces enjeux, la commission a introduit plus de souplesse pour accompagner une relance du don croisé compatible avec les exigences liées à cette procédure complexe. Elle a également affirmé un « statut de donneur », préconisé par le Comité consultatif national d'éthique comme par les associations. Je souhaite que le Gouvernement puisse se saisir de ce cadre comme d'une opportunité de mieux valoriser, même symboliquement, ce geste altruiste et civique qu'est le don d'organes.

ou d'exclure du prélèvement les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection avec représentation à la personne. Suivant cette même logique, la commission a ouvert le don du sang dès l'âge de 17 ans, afin de permettre aux jeunes de contribuer à la solidarité nationale par ce geste citoyen. Le projet de loi apporte en outre des clarifications bienvenues à l'encadrement de l'interruption de grossesse pour motif médical et des réductions embryonnaires ou foetales. Sur le sujet de l'interruption médicale de grossesse, la commission spéciale n'a pas jugé nécessaire de prévoir une clause de conscience spécifique des professionnels de santé, dès lors qu'une clause de conscience générale leur permet déjà de ne pas accomplir un acte contraire à leurs convictions. Enfin, la commission spéciale a adopté, en y apportant des améliorations, le dispositif proposé par l'Assemblée nationale sur la prise en charge des enfants présentant une variation du développement génital par les centres de référence. Elle a notamment soumis le diagnostic et la prise en charge de ces enfants à un référentiel de bonnes pratiques, arrêté par la Haute Autorité de santé en concertation avec les associations de patients. Telles sont les principales observations sur les articles du projet de loi dont je suis le rapporteur et que la commission spéciale vous demande d'adopter. J'ajoute à ces considérations ma conviction que ce projet de loi nous offre une opportunité, celle de démontrer que le progrès de la connaissance peut être, est bénéfique à notre population. L'enjeu est de poser le cadre dans lequel la connaissance scientifique doit progresser, et certainement pas de l'empêcher. Avoir conscience, identifier les dérives possibles et instituer les garde-fous nécessaires relèvent du rôle irremplaçable du législateur. Nous légiférons dans un monde ouvert : notre responsabilité n'en est que plus complexe. Ayons ensemble la volonté commune de dépasser ces obstacles dans le consensus tant nous savons que l'obscurantisme est simplement le fils de l'ignorance et de l'intolérance. La parole

les clivages traditionnels ne tiennent plus. Tous les groupes politiques ont d'ailleurs renoncé à donner une consigne de vote, pratique que le groupe du RDSE expérimente régulièrement. La France a fait le choix de confier aux représentants du peuple, et donc au peuple, les décisions en matière de bioéthique. C'est le peuple qui tranche sur le permis et l'interdit face à des progrès scientifiques qui font que la médecine ne se contente plus de soigner les malades.

c'est à nous, en tant que représentants du peuple, de nous prononcer sur notre propre conflit de valeurs, en gardant toujours à l'esprit l'intérêt général, qui n'est jamais la somme des intérêts particuliers. Ces dilemmes éthiques se résolvent non par l'absolutisme d'une valeur sur les autres, mais par la recherche de solutions qui prennent en compte les avancées de la science et de la société. En cela, je le disais, ce projet de loi ne ressemble à aucun autre. Il pose une question simple dont la réponse est complexe est-ce que la société veut ce que la science peut ? En d'autres termes, est-ce que cela doit être autorisé parce que cela est possible ? Considérant, comme le dit si bien Jean Leonetti, qu'il est important de continuer à énoncer l'interdit, je m'efforcerai de vous présenter ma position sur les grandes mesures de ce texte, hormis celles qui concernent le don d'organes sur lesquelles mon collègue Jean-Pierre Corbisez se prononcera. Bien qu'étant cheffe de file de mon groupe, je m'astreindrai à parler en mon nom propre, afin de laisser à mes collègues le soin de se faire leur propre avis au fil des discussions.

loi ne contient pas. La gestation pour autrui, l'eugénisme et les chimères ne figurent pas dans ce texte, et rien ne permet d'affirmer que ses dispositions ouvrent une quelconque porte à leur légalisation.

effet, le législateur a mis en place un dispositif efficace qui permet soit d'interdire une technique, soit de l'autoriser dans un cadre qui limite les risques et garantit les évaluations.

projet de loi. Les enfants issus d'une GPA à l'étranger existent : nous ne pouvons pas les ignorer. Considérant qu'il faut d'abord les protéger, j'ai déposé un amendement de suppression de l'article 4 relatif à la transcription de l'acte de naissance des enfants nés d'une GPA à l'étranger l'enfant n'est pas responsable de son mode de procréation et ne doit pas en être pénalisé. J'en viens maintenant à la question qui a occupé et qui occupera une bonne partie de nos discussions : l'extension de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes célibataires- je préfère ce terme à celui de femmes « seules » qui reflète, à mon sens, un jugement de valeur discutable. D'abord, sur la forme, je suis d'avis que cette mesure aurait dû faire l'objet d'une loi à part, une loi sociétale à l'instar de celle sur le mariage pour tous.

Cela étant, j'ai abordé ce sujet comme j'essaie d'aborder toutes les questions sociétales : avec humilité, pragmatisme, progressisme et humanisme. Tout en gardant à l'esprit l'intérêt de l'enfant, souvent brandi avec force par les opposants à la réforme, je suis convaincue que, correctement régulée, la technologie renforcera le seul modèle familial qui prévaut, celui qui est fondé sur l'amour. La légalisation du mariage pour tous avait fait craindre à certains la destruction d'un modèle familial classique, fondé sur un couple hétérosexuel marié et des enfants. cela fait bien longtemps que ce modèle a été rejoint par d'autres. Il est nécessaire aujourd'hui de reconnaître la diversité des configurations familiales qui composent notre société. Rappelons d'ailleurs que les célibataires peuvent adopter depuis 1996 et qu'il est interdit de leur refuser l'agrément pour ce seul motif. Dans le cas de l'adoption, comme dans le cas de la PMA, il s'agit de procédures longues qui nécessitent une réflexion mûrie, de la patience et de la détermination. On parle d'enfants attendus, désirés, parfois viscéralement. On parle de fonder la famille sur une base plus solide que la seule procréation, qui est un acte biologique, tandis que la parentalité est un acte social et affectif. Pour ma part, vous l'aurez compris, je suis résolument convaincue de l'intérêt d'étendre la PMA à toutes les femmes, je défendrai deux convictions lors de l'examen de l'article 1. Tout d'abord, pour une question d'égalité, il me paraît essentiel de garantir à toutes les femmes le remboursement de la PMA, seule condition de l'existence d'un droit réel, non soumis à des critères financiers.

Ensuite, dans une perspective humaniste et parce que la situation actuelle n'est pas acceptable, je défendrai un amendement permettant aux femmes de bénéficier du transfert des embryons issus d'une fécondation en cas de décès de leur conjoint en cours de procédure. Aujourd'hui, ces embryons sont soit détruits, soit donnés à un autre couple. Demain, la femme, elle-même veuve, pourra bénéficier d'une PMA avec

Sur les dons de gamètes, les débats sont tout aussi complexes. Si l'on comprend naturellement le besoin des enfants nés d'une PMA avec donneur de connaître leurs origines, nous sommes nombreux à craindre une forte baisse des dons alors que ceux-ci ne permettent déjà pas de répondre à toutes les demandes. Certains membres de mon groupe soutiendront un amendement visant à revenir au droit actuel, c'est-à-dire à l'anonymat du donneur. Pour ma part, je suis plutôt favorable au compromis trouvé en commission, qui prévoit que l'agence sollicite l'accord du donneur au moment de la demande de l'enfant, ce qui permet de respecter le désir de l'enfant et la vie privée du donneur, tout en préservant le stock de gamètes Sur d'autres sujets, je m'associe à l'excellent travail des rapporteurs. Je ne défendrai donc aucun amendement sur l'extension à titre dérogatoire de la recherche sur le développement des embryons jusqu'à l'autorisation à titre expérimental du diagnostic préimplantatoire pour la recherche d'aneuploïdies en vue d'améliorer la prise en charge des femmes en AMP et le taux de réussite des fécondations, sur sur la suppression de la double clause de conscience spécifique à l'interruption médicale de grossesse, ou encore sur la prise en charge des enfants présentant une variation du développement génital, dans la mesure où il est nécessaire d'optimiser la prise en charge actuelle. Au-delà de mes convictions, qui me poussent à soutenir la plupart des mesures du texte initial, je suis convaincue qu'il faut laisser plus de liberté aux professionnels de santé et à nos concitoyens, en respectant la volonté, les désirs et la capacité de chacun à décider en responsabilité. Je salue en ce sens les Je salue en ce sens les avancées obtenues en commission : elles permettent d'introduire des critères plus souples sur l'âge en cas d'autoconservation des ovocytes et de PMA. Comme je l'ai souvent dit, la reconnaissance tardive de maladies telles que l'endométriose ainsi que le défaut d'information des patientes doivent nous encourager à faire davantage, notamment en termes de préservation de la fertilité. Je terminerai en rappelant que, sans une politique familiale volontaire et une meilleure prise en compte de la grossesse des femmes dans le monde du travail et dans la société, toutes ces bonnes intentions pourraient demeurer vaines. La parole

Face à ces évolutions, celles des dernières années et celles à venir, le projet de loi relatif à la bioéthique soumis à notre examen comporte des avancées majeures et un cadre nécessaire à leur inscription dans ce contexte sociétal. Avant d'évoquer dans le détail certaines dispositions du texte de notre commission spéciale, je tiens à rappeler l'un des engagements forts d'Emmanuel Macron, alors candidat à la présidence de la République, concernant, en particulier, l'une des mesures phares de ce projet de loi celui de reconnaître et de permettre à chacun de vivre sa vie de couple et ses responsabilités parentales et, pour ce faire, d'inclure pleinement l'ensemble des familles du pays, de plus en plus diverses, et ainsi de tenir compte du fait qu'il n'y a bel et bien pas un modèle unique qui représenterait la « vraie » famille. Dit ainsi, cela paraît assez simple : « On le dit. On le fait. » Il n'en est rien. La volonté du Gouvernement depuis le début des travaux a été de tenir une ligne d'équilibre, sans brusquer les débats. il n'est nullement question de changer de boussole ni de rompre avec les trois principes qui fondent les lois bioéthiques françaises : la dignité, la liberté et la solidarité. Dans un esprit constructif et respectueux des convictions de chacun, le texte s'est notamment appuyé sur les travaux des États généraux de la bioéthique de 2018, organisés par le Comité consultatif national d'éthique. Cette institution est est des plus précieuses, tant sur le fond que pour son savoir-faire dans l'organisation de la concertation autour de ces sujets. Le texte que nous examinons aujourd'hui est issu des travaux de notre commission spéciale. Je tiens avant tout à saluer le travail de son président et de nos quatre rapporteurs. Les auditions et les débats au sein de la commission, d'une grande qualité, se sont tenus dans le respect de la légitimité des divers points de vue exprimés. Je souhaite également préciser que, sur bien sur bien des sujets abordés, les discussions au sein de notre groupe La République En Marche ont vu émerger des points de vue le plus souvent convergents, mais pas toujours. Loin de chercher à constituer un bloc monolithique, nous avons au contraire tenté, et je l'espère, réussi à laisser suffisamment de place au débat. J'insiste sur cette nécessité de prendre en compte les avis et sensibilités de chacun, tout en appréciant nos débats apaisés. C'est un cheminement commun qui nous a permis de mûrir nos réflexions. Notre groupe soutiendra pour l'essentiel les évolutions prévues par le projet de loi initial, ce qui nous amènera, sur certains points, à soutenir des amendements de suppression ou de réécriture du texte issu de la commission. Dans un esprit constructif, j'évoquerai en premier lieu les points d'accord avec notre commission spéciale- et ils sont nombreux. favorables au principe de l'ouverture aux couples de femmes et aux femmes seules de la procréation médicalement assistée, ainsi qu'à l'ouverture du droit à l'accès aux données non identifiantes pour les enfants issus de dons et aux données identifiantes sous condition, par l'intermédiaire d'une commission que nous souhaitons rétablir. Nous soutenons l'autoconservation des gamètes, afin de tenir compte des problèmes d'infertilité et des évolutions sociétales. Nous défendons également l'ouverture du don de sang aux mineurs de 17 ans et majeurs sous protection juridique, mesure issue de l'amendement de notre rapporteur Bernard Jomier. Sur le plan de la recherche et des moyens autorisés pour la promouvoir, pour la promouvoir, plusieurs dispositions recueillent notre soutien, comme la distinction et le contenu des régimes juridiques de la recherche sur les cellules embryonnaires et de celle sur les embryons. Je m'associe également à l'idée d'une extension du recueil et de la conservation des dons de gamètes aux centres privés. De même, je soutiendrai le nouvel article 19 autorisant,

notre groupe approuve la suppression de la clause de conscience spécifique des professionnels de santé en matière d'interruption médicale de grossesse. Autre point d'accord avec notre commission spéciale, la suppression de la création de délégations parlementaires à la bioéthique, disposition que l'Assemblée nationale avait introduite dans le texte. J'évoquerai maintenant nos points de désaccord avec la commission spéciale, notamment l'article 1qui occupera une grande partie de nos débats.

de dignité et de solidarité. À nos yeux, la conciliation entre ces trois principes qu'a réalisée la commission n'est ni satisfaisante ni équilibrée, ce qui légitime nos amendements. Le premier vise à revenir au sens initial du projet de loi, c'est-à-dire l'extension de la PMA en réponse aux projets parentaux, et ce sans distinction, sans retenir un critère pathologique

de toute prise en charge par la sécurité sociale. L'esprit de ce texte est de trouver des solutions aux difficultés rencontrées par ces personnes pour réaliser leur projet parental, désormais aussi légitime que tout autre. Dès lors, nous nous refuserons toujours, comme nous y conduit le texte de la commission, à distinguer les situations selon des critères d'orientation sexuelle ou de composition des ménages, les bons projets parentaux qui méritent le soutien de la solidarité nationale des « moins bons » qui, eux, ne seraient pas pris en charge. Nous voulons encourager l'ensemble des projets parentaux ; nous ne voulons en juger aucun. Ce n'est ni notre vision de la solidarité ni notre conception de la famille. Par ailleurs, il nous semble contradictoire et injuste de maintenir l'interdiction de la procréation, alors qu'est offerte aux femmes seules la possibilité d'accéder à ces techniques. Face à de tels cas, très rares, nous défendrons un amendement pour éviter un double deuil aux femmes concernées. S'agissant du droit d'accès à leurs origines des personnes issues d'un don, un point clé du texte, nous partageons la volonté de rompre avec la culture du secret et de faire progresser la transparence sur ces sujets au sein des foyers. Nous pensons que le texte peut aller plus loin. Aussi, nous vous proposerons un amendement pour objet d'informer les receveurs de dons de gamètes ou d'embryons sur le besoin de transparence et d'information des enfants.

la dimension psychologique et sociale de l'évaluation par l'équipe pluridisciplinaire et le rappel des possibilités d'adoption lors de leur parcours. Sur ce point, nous ne doutons pas que les personnes s'inscrivant dans un protocole aussi lourd

Enfin, je soutiendrai avec plusieurs de mes collègues un amendement visant à ce que l'établissement de la filiation d'un enfant à l'égard des deux femmes d'un couple ne se traduise pas dans l'acte de naissance par une rédaction spécifique et, donc, distinctement identifiable. Je conclurai par un constat. Le corps des femmes a trop souvent fait l'objet de débats, comme s'il s'agissait d'un bien public devant être contrôlé, encadré. Aujourd'hui, nous allons légiférer une nouvelle fois sur le sujet, mais il s'agit là de permettre aux femmes, sans distinction, d'accéder à la procréation médicalement assistée et de former des projets de parentalité dans le respect de la dignité, de la liberté, de la solidarité et de l'intérêt supérieur de l'enfant. En ces instants, chacune et chacun d'entre nous a à l'esprit, quelles que soient ses convictions, le poids de la responsabilité du législateur. Écoutant Montesquieu, certains préféreraient peut-être ne toucher aux lois « que d'une main tremblante ». À titre personnel, j'ai pleine confiance dans la nature et la qualité des échanges que nous aurons dans cet hémicycle. Ils nous conduiront, je le souhaite, à faire les bons choix pour l'avenir. Avec discernement, mais sans trembler ! La parole

qui n'a pas été tant modifié que cela. Qui s'en étonnera ? Sans constance et sans conviction, par crainte d'apparaître ringards, vous cédez à l'air du temps, à la mode, la mode, qui n'est pourtant que l'expression de l'éphémère. Par ce sabordage, par cette capitulation devant ceux qui ne sont assurément pas les plus nombreux, mais qui crient sans doute le plus fort, notre pays bascule dans la libéralisation mondialisée de la procréation, ouverte au marché et aux puissances de l'argent. Le droit l'enfant s'efface au profit, c'est le cas de le dire, du droit l'enfant ! L'Académie nationale de médecine parle d'une « rupture anthropologique majeure » et, ce dimanche encore, des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour s'opposer à cette nouvelle régression. Puisque l'humain et la vie n'échappent plus au législateur et sont sacrifiés sur l'autel de l'idéologie et du tout-mercantilisme, nous entrons dans le totalitarisme sociétal où l'enfant est non plus un don mais un achat, non plus le fruit de l'amour entre un homme et une femme, non plus celui d'une mère et d'un père, mais un produit de consommation amputé, privé de l'indispensable paternité. Où sont la hauteur de vue et le débat ? En matière de bioéthique, comme en bien d'autres domaines, nous assistons à une caricature de la démocratie représentative. Cela mérite une vraie remise en question de la part de chacun d'entre nous, car ce sujet ne concerne aucun parti politique, aucune chapelle, aucun partisan. Il fait appel avant tout à l'éthique. Mais de quelle éthique s'agit-il ici ? À ce qui semble être votre éthique normative, reposant sur l'égalitarisme et l'utilitarisme et dont le but prétendu serait la justice sociale, j'oppose et propose l'éthique appliquée, reposant, elle, sur la déontologie, sur la conformité à notre devoir. Or notre devoir, mes chers collègues, c'est de penser à l'intérêt de l'enfant, plutôt qu'au désir de l'adulte, qui a manifestement perdu la raison. Dès lors, ce qui est scientifiquement possible n'est pas forcément éthiquement acceptable. À force d'être en marche perpétuelle, à force de ne plus être rattachés à rien, de n'avoir plus aucun repère, auriez-vous perdu à ce point l'esprit en traitant de l'éthique de l'homme et de la vie comme vous traiteriez du plus anecdotique des textes de nos lois ? Vous êtes en train de détruire le dernier et le plus important pilier que l'on retrouve dans toutes les civilisations, celui du droit de l'enfant à naître au sein d'une famille gouvernée et protégée par sa mère par son père. Sous couvert de liberté et d'égalité, nous piétinons la fraternité, l'altérité et la paternité. Il s'agit là d'avoir une réflexion anthropologique de fond, et non d'assister à une énième succession de polémiques et de « coups » dits progressistes à visée électorale.

par une remise en question des dérives de ceux qui ont mené la révolution de mai 68, demandé et obtenu de « jouir sans entraves ». Ne serons-nous pas frappés, demain, par une remise en question sur la manière dont on a menti à des enfants sur leur filiation biologique, sur les circonstances légales qui auront permis, progressivement, la marchandisation des corps ? Votre société faussement « inclusive » est en réalité une société oppressive, voire d'exclusion- exclusion du père, fragilisant l'enfant. Le droit à la vie, à la dignité et au respect est anéanti par un eugénisme rêvant d'un monde où l'on sélectionne ceux qui ont le droit de vivre et dans lequel le handicap est reçu comme une tare à supprimer. Il est moche, votre mythe du progrès Notre responsabilité est de permettre aux enfants de France de venir au monde et de grandir dans des conditions favorables, dans des familles où l'altérité permet la stabilité, où la complémentarité permet l'épanouissement, où l'égalité entre hommes et femmes peut enfin s'appliquer. Par ailleurs, après les OGM, les manipulations de gamètes et d'embryons permettront aux laboratoires de proposer des HGM, des humains génétiquement modifiés. Face à cette découverte scientifique, qui est une folie sur le plan de l'éthique, nous sommes le dernier rempart Réalise-t-on ce qu'est la FIV, fécondation, ? La congélation d'un embryon, permettant qu'un enfant puisse naître en étant biologiquement orphelin, est une atteinte grave à l'enfant lui-même ! De ce progrès-là, nous ne voulons pas Replongeant dans nos racines grecques, nous comprenons l'et la démesure comme un orgueil destructeur. Voici revenu le temps des limites ! C'est pourquoi, comme à notre nation nous proposons des limites géographiques et comme dans le domaine de l'écologie nous proposons le localisme, sur le plan éthique et anthropologique nous vous exhortons à adopter le principe de précaution, de préservation, en refusant en conscience ce texte de loi qui ouvre la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules. Mes chers collègues, ne cédez pas aux ayatollahs d'une société sans racines, sans pères et sans repères ! À la société de l'envie, préférons toujours la société de la vie

pour la qualité de notre travail. Les nombreuses auditions menées ont permis de nous éclairer sur un certain nombre de sujets. Certains étaient complexes, d'autres sensibles, mais toutes ces auditions se sont déroulées dans un climat serein. Je remercie également Mmes les ministres d'avoir organisé des séminaires ouverts à tous les parlementaires. La révision des lois de bioéthique nous confère une grande responsabilité sur l'avenir du genre humain, sur les limites que nous voulons poser pour définir ce qui est scientifiquement et techniquement possible, d'une part, et éthiquement souhaitable, d'autre part, pour ne pas dénaturer l'espèce humaine, pour ne pas « marchandiser » le vivant. Toute avancée technique ne constitue pas en elle-même un progrès, et c'est à nous, en tant que législateurs, de mettre des garde-fous. Il n'est pas toujours simple de se projeter dans l'exploration d'un monde inconnu, rendu perceptible par l'évolution des connaissances et des technologies, de dépasser certaines frontières sans s'affranchir des principes fondant notre société. Comment continuer à avancer vers l'émancipation et le progrès sans basculer vers une dystopie, telle que décrite par Aldous Huxley dans ? Parlementaire communiste, je suis particulièrement sensible à ces deux aspects et résolument déterminée à faire obstacle aux forces financières et marchandes qui veulent faire voler en éclat notre modèle social et éthique. J'en viens au texte lui-même, en centrant mon propos sur les droits humains, Éliane Assassi intervenant également pour notre groupe. Ouvrir la PMA à toutes les femmes, qu'elles soient en couple avec une autre femme ou seules, est pour nous un acte fort, un réel pas en faveur en faveur de l'égalité. D'ailleurs, nous avions régulièrement déposé des amendements allant en ce sens sur des textes précédents. C'est une avancée attendue, promise depuis des années, enfin obtenue après une longue bataille pour mettre fin à une discrimination, fondée notamment sur l'orientation sexuelle. En ouvrant la PMA aux couples lesbiens, nous allons mettre fin à une inégalité hypocrite. Hypocrite, car cette pratique est autorisée dans plusieurs pays voisins et de nombreuses femmes françaises se rendent chaque année à l'étranger pour pouvoir fonder une famille. Ainsi, à la discrimination reposant sur l'orientation sexuelle, s'en ajoutait une autre fondée sur l'argent, au regard du coût d'une PMA à l'étranger. Hypocrite, car depuis 2013 et la loi sur le mariage pour toutes et tous, alors qu'il est possible pour les couples de même sexe d'adopter et, donc, d'être parents- cela reste néanmoins très difficile -, il n'était pas possible pour les couples de femmes d'avoir accès à la PMA. Cet élargissement du droit à la PMA, dans un contexte où l'homophobie est encore très présente en France, peut donc contribuer à un peu plus d'égalité, en mettant fin à une sorte d'homophobie institutionnalisée. Comme l'a très justement dit l'une des représentantes d'associations LGBT que nous avons auditionnées, « la République doit protéger de la même façon tous les enfants L'article 1 de ce projet de loi est donc majeur. Au sein du groupe CRCE, nous serions heureux et heureuses de pouvoir le voter. Mais c'est à la condition que l'amendement de la rapporteure Muriel Jourda, accepté en commission, soit supprimé. N'est-il pas une façon détournée d'exclure encore et toujours les couples de femmes et les femmes seules, puisque le remboursement de la PMA serait conditionné par le caractère pathologique ? J'en viens à présent à l'autre grande avancée de ce texte : la levée de l'anonymat en cas de recours à l'AMP. Là encore, cela répond à une demande légitime, de la part d'enfants nés par don, d'avoir accès à leurs origines, s'ils le souhaitent, à leur majorité. Nous avons entendu la souffrance qu'expriment un certain nombre d'entre eux d'être confrontés à un vide dans leur histoire personnelle. Ils pourront désormais le combler, s'ils en ressentent le besoin. Dire cela, ce n'est pas dire que le géniteur est un père, un parent. Bien au contraire ! Dire cela, c'est reconnaître que, dans bien des familles hétérosexuelles, le silence, le tabou autour d'une conception par par PMA peuvent être douloureux si l'enfant ne connaît pas toute son histoire. Pour autant, et c'est essentiel, l'un de nos principes éthiques fondamentaux est garanti et préservé, puisque l'anonymat restera entre le donneur et le couple receveur. Par ailleurs, nous saluons le fait que le texte fasse évoluer notre législation en faveur d'autres dons, que ce soit le don croisé d'organes pour les greffes rénales ou le don d'organes, de tissus et de cellules des majeurs En leur permettant de donner leurs organes, à des fins scientifiques et médicales, et ainsi d'entrer dans le droit commun, nous allons vers une meilleure reconnaissance des majeurs protégés, tout en posant une limite éthique pour le prélèvement, sur adoption d'un amendement du rapporteur Bernard

plus au regard de l'évolution des techniques médicales. J'entends bien les craintes exprimées par plusieurs de mes collègues sur les risques de dérive, de sélection, pour ne pas dire d'eugénisme. Mais je crois que la définition proposée ne nous conduit pas vers de tels écueils, tout en évitant à des femmes, à des couples déjà engagés dans une procédure lourde et difficile de connaître plus de plus de complications en termes de santé ou de multiplier les fausses couches. Là aussi, il me semble que nous sommes parvenus à un équilibre entre avancées scientifiques, droits nouveaux et principes éthiques garantis. Je ne pourrais pas terminer mon intervention sans effleurer la problématique des enfants présentant une variation du développement sexuel, qui ne figurait pas dans le projet de loi initial. Nous avions déjà eu l'occasion, dans le cadre de la délégation aux droits des femmes, de nous intéresser à ce sujet et de comprendre les difficultés de ces enfants, notamment de celles et ceux qui ont été opérés et à qui a été attribué attribué un sexe ne correspondant pas à leur genre. Même si, aujourd'hui, les opérations à la naissance sont de moins en moins pratiquées, nous pensons, au groupe CRCE, qu'il faut aller plus loin et les interdire, sauf en cas de nécessité médicale. texte, effectivement, a pu nous bousculer dans nos certitudes, nous plonger dans un futur fantasmatique parfois proche de la science-fiction, tant les évolutions médicales et scientifiques sont rapides, mais également dans un futur inquiétant,

la société et la science évoluent. Il semble normal que la loi évolue, elle aussi, pour accompagner ces changements. Pourtant, notre rôle n'est pas d'autoriser tout ce que la technique permet de réaliser. Nous devons sélectionner, parmi le champ des possibles, ce qui est souhaitable. C'est l'essence même de la politique ! « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », écrivait l'auteur de voilà presque 500 ans. Aussi, l'exercice de révision des lois de bioéthique est toujours un exercice périlleux, qui engage la responsabilité et la conscience de chacun d'entre nous. Nous avons chacun nos convictions, et mon groupe respecte l'ensemble des sensibilités qu'il représente. Aussi, je m'exprimerai de façon personnelle et j'ai bien conscience de ne pas représenter la majorité des convictions de mon groupe, ce dernier restant très partagé sur ces questions. Les valeurs que je défends me semblent être celles d'un humanisme éclairé, animé par une vision pragmatique. Je tiens tout d'abord à féliciter et remercier le président et les rapporteurs de la commission spéciale pour leur travail de grande qualité. Le texte adopté par la commission est le fruit d'un travail collectif, éclairé par les nombreuses personnes très compétentes qui ont été auditionnées. À l'article 1, je suis favorable à l'ouverture de la procréation médicalement assistée pour les femmes seules-

autant, même si certains peuvent penser que ce n'est pas égalitaire, il ne revient pas à l'assurance maladie de prendre en charge cette technique lorsqu'elle n'est pas motivée par un critère médical. Je suis donc favorable aux amendements adoptés par la commission spéciale visant à limiter la prise en charge de l'AMP par la solidarité nationale aux couples médicalement infertiles. Je pense également que nous devons préserver le dispositif d'évaluation médicale et psychologique des futurs parents ou de la future mère comme condition préalable à l'AMP. Par ailleurs, la gestation pour autrui représente une ligne rouge en matière de bioéthique, que nous ne devons pas franchir. Les avancées sur la PMA pour les couples de femmes ne sauraient constituer un premier pas en direction de la GPA pour les couples d'hommes. Le ventre d'une femme n'est pas commercialisable- selon les termes mêmes de la Constitution de 1793 -et la reproduction n'est pas un nouveau facteur de production. Je suis donc opposé à tout fléchissement de la législation en direction de la GPA. Je suis favorable au maintien de l'anonymat des donneurs de gamètes, lorsque ces derniers ne souhaitent pas être identifiés par les enfants issus de leurs dons, comme je suis favorable à la communication systématique des données non identifiantes à ces mêmes enfants, lorsqu'ils en font la demande à leur majorité. J'avais proposé un amendement de réécriture de l'article 3 en ce sens. Je remercie la commission spéciale de l'avoir repris et intégré dans le texte, conformément à l'avis du Conseil d'État. Je considère que nous ne pouvons pas, dans un même texte, augmenter le nombre de demandeurs de gamètes en ouvrant l'accès à l'AMP, tout tout en ne respectant pas complètement l'anonymat des donneurs qui le souhaitent, ces derniers, je le rappelle, n'étant pas rémunérés en France. Je pense aussi qu'il est important de maintenir le consentement du conjoint du donneur, si ce dernier est en couple, comme le prévoit la législation actuelle et bien qu'elle soit parfois contournée. Actuellement, les AMP avec tiers donneur ne représentent que 4 % des pratiques réalisées, mais ce chiffre est appelé à augmenter avec l'ouverture de cette pratique aux couples de femmes et aux femmes seules. L'accès à l'AMP est une question difficile. Nous aurons l'occasion d'en débattre en séance. Je réserve mon vote sur cette question, bien que je sois plutôt favorable, dans la mesure où la femme aurait de toute façon la possibilité d'effectuer une AMP en tant que femme seule par la suite. Je suis favorable à l'autorisation de l'autoconservation des gamètes à des fins de prévention de l'infertilité, ainsi que le prévoit l'article 2 du projet de loi. La commission a assoupli les conditions d'âge pour effectuer ces autoconservations. Il me semble que cela représente une avancée louable pour les patients et les patientes exposés à un risque particulier d'infertilité. Encore une fois, je félicite la commission spéciale d'avoir adopté un amendement visant à élargir la conservation des gamètes

favorable au diagnostic préimplantatoire élargi à la recherche d'anomalies chromosomiques au-delà des seules anomalies préalablement identifiées dans la famille. Comme l'a indiqué

J'émettrai des réserves quant aux expérimentations sur les embryons chimériques animal-homme. La commission a souhaité encadrer, à juste titre, cette possibilité, en prévoyant une limite de 50 % de cellules pluripotentes pluripotentes induites humaines dans un embryon d'animal, sans évoluer, bien sûr, vers la parturition. Je suis favorable à l'interdiction d'expérimentations visant à introduire des cellules souches embryonnaires humaines dans un embryon animal, en accord avec la commission spéciale du Sénat. Le retour à un régime d'autorisation pour ces recherches bien spécifiques pourrait être préférable à une simple déclaration auprès de l'Agence de la biomédecine. Par ailleurs, le régime dérogatoire est nécessaire pour améliorer les recherches et encourager le progrès

ectodermiques apparaissent, préfigurant l'élaboration du cerveau. Je suis favorable à l'abaissement à 17 ans de l'âge légal pour pouvoir donner du sang, tout comme à la création d'un statut, honorifique, de donneur d'organe. Madame le ministre, je souhaite aussi attirer votre attention sur la prévention du trafic d'organes humains ; il me semble que la France n'a pas encore ratifié le traité de Saint-Jacques-de-Compostelle à ce sujet, contrairement à bon nombre de nos voisins. Je défendrai des amendements pour sécuriser et favoriser les dons d'organes. En effet, 100 à 200 personnes meurent en France faute de greffons. Aussi, je proposerai la création d'une liste prioritaire de greffe de rein pour les donneurs de leur vivant qui auraient, par la suite, un besoin vital d'un greffon. Cette situation est, bien sûr, extrêmement rare, mais elle constitue souvent un frein psychologique au don de rein. Je proposerai également un amendement visant à renforcer

amendé par la commission spéciale, apporte des avancées que je considère comme positives pour notre pays. Il permet d'adapter, dans un sens pragmatique et utile, le développement de la biomédecine à l'évolution sociétale. La

ce texte échappe aux classifications routinières ! Sylviane Agacinski, Michel Onfray, Alexis Escudero, mais aussi José Bové, Marie-Jo Bonnet et d'autres encore ne viennent pas de la même planète politique que la mienne.

figure au frontispice de tout l'édifice juridique de la bioéthique. La dignité, c'est-à-dire la fragilité. La fragilité, donc la fraternité

nous voulons à tout prix la fraternité des coeurs, il ferme les yeux, souvent, trop souvent, sur la marchandisation des corps. Quand nous proclamons

elle exerce une formidable pression sur nos juges, sur le législateur que nous sommes individuellement et collectivement. Souvent

en dépit de la volonté du peuple français. Ce n'est pas ma conception de la souveraineté populaire ! Qu'est-ce qui m'autorise à évoquer un alignement, un rapprochement entre deux modèles ?

tant que président d'un département d'un service d'aide sociale à l'enfance. Qui ne sait pas que les situations de monoparentalité augmentent les risques de fragilité pour le parent isolé

nous avons à accomplir une oeuvre législative difficile, qui nous interroge sur le vivant, sur nos règles en société, sur notre conception de la société et sur nos valeurs. Le rapport de l'homme avec ses inventions compte parmi les grands risques », disait, il fut un temps, un membre du Comité consultatif national d'éthique. L'histoire, la littérature, le théâtre, l'opéra nous racontent ce conflit entre la folie des savants et les dangers pour l'humanité. Méphisto n'est pas loin, qui veut entraîner Faust dans des endroits dangereux

Il est légitime que nous nous dotions d'une loi nationale, même si nous vivons dans un monde sans frontières et sans règles internationales.

Pour autant, si notre législation nationale est légitime, et elle doit exister, parce que nous sommes au coeur de la République, elle ne peut pas ne pas tenir compte de l'accès de nos concitoyens à d'autres sphères de règles juridiques ni à des réalités que des réalités que l'ère numérique a créées. C'est d'ailleurs en ce sens que notre rapporteur a proposé d'accepter les tests génétiques à visée généalogique, en déclarant qu'il valait mieux protéger nos concitoyens que de les laisser enfermés auprès de sociétés étrangères, avec moins de protections. Cette législation nationale est légitime et doit être inspirée par des valeurs qui nous sont propres et qui ne sont pas forcément celles de tous les pays européens.

et essentiellement la non-patrimonialité du corps humain. C'est la gratuité du don qui justifie d'ailleurs un amendement de la commission visant

C'est pourquoi personne n'a proposé, ici, un amendement légalisant la GPA. La question des droits de l'enfant est un autre sujet. Le désir d'enfant est légitime, mais il n'ouvre en aucun cas le droit à l'enfant.

Ces principes sont des boussoles qui nous interrogent face aux progrès scientifiques. Ces interrogations, comme l'a dit le précédent orateur, transcendent nos groupes politiques.

que d'autoriser la création d'une filiation née d'un projet parental assisté, parce que la médecine le permet, dans des limites que nous devons fixer. Sur les titres II, III et IV, notre commission, madame la ministre, a été moins stricte que le texte émanant de l'Assemblée nationale, sur lequel nous avons bien compris, en entendant quelles étaient vos lignes rouges, que vous aviez largement pesé, dans cette majorité de l'Assemblée, pour ne pas accepter, s'agissant notamment de sujets qui avaient reçu des avis conformes de la part du Comité consultatif national d'éthique.

Jean Jaurès : « Les progrès de l'humanité se mesurent aux concessions que la folie des sages fait à la sagesse des fous. » Si les savants sont des fous,

d'opérer cette synthèse entre la sagesse des fous et la folie des sages, et nous permettrons à l'humanité de faire un progrès sans bouleverser nos valeurs

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, quelle fierté de vivre dans un pays qui a inscrit la bioéthique dans son histoire législative ! Et le Sénat n'y est pas étranger

Mais, depuis 1994, saluons l'intérêt que suscitent ces débats avec l'émergence de nombreux acteurs : l'Agence de la biomédecine, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et, bien sûr, le Comité consultatif national d'éthique- sans parler des comités d'éthique qui existent partout où les questions se posent. Eh oui, on peut le dire, notre démocratie respire et inspire ! La société fait débat et le débat fait société. Pour tout dire, peut-être comme beaucoup d'entre vous, je doute. Je redoutais aussi ce texte. Est-ce une faiblesse, est-ce une force ? Là n'est pas la question. Sur ces questions de bioéthique, j'avoue, je partais avec un capital de doute énorme. Aussi, j'ai participé activement aux travaux de la commission spéciale. Prendre ses responsabilités, c'est mieux cerner les enjeux. Prendre des décisions, c'est comprendre la réalité, sa perpétuelle évolution et les questions sociétales qui s'y rattachent. Je tiens à saluer mes collègues de la commission spéciale pour l'infini respect qu'ils ont porté à la parole et aux convictions de chacun pendant nos travaux. Empathie, respect et humilité, telles sont mes boussoles pour l'examen de ce texte. Venons-en maintenant au contenu de ce projet de loi de bioéthique. L'article 1 tend à éclipser les dizaines d'articles qui lui succèdent, alors qu'ils auront,, un impact tout aussi important sur la société : l'autoconservation des gamètes, l'utilisation de l'intelligence artificielle, des diagnostics prénataux, la favorisation des dons croisés, et j'en passe. Il vise à élargir l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes célibataires, comme dit Véronique Guillotin. J'y suis favorable. Cela relève beaucoup de l'intime, de notre éducation et de nos parcours personnels mon choix m'appartient, il n'est en aucune façon celui de chacun des collègues de mon groupe ; chacun a son cheminement, chacun a ses convictions, et tout choix est respectable. L'idée que ce débat aurait pu être séparé de l'ensemble de la loi de bioéthique est à mon avis une échappatoire. En réalité, l'AMP a été inscrite dans la loi de 1994. Il est donc tout naturel que nous en débattions de nouveau lors de cette révision. Revient souvent l'argument que d'être élevé par un couple de femmes ou une femme célibataire serait nier l'importance de l'altérité. La comparaison un peu forte, mais mon expérience auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de mon département m'apporte malheureusement souvent la preuve que l'altérité n'est pas toujours heureuse. Par ailleurs, nous observons que la famille est aujourd'hui multiforme. Le nombre de familles monoparentales ne démontre pas non plus une éducation défectueuse ou altérée. L'établissement d'un projet parental ne garantit sans doute pas une excellence dans la future parentalité, mais il assure, je le crois, une intention réfléchie et construite.

en introduisant le critère d'infertilité ou de non-transmission d'une maladie d'une particulière gravité aux couples hétérosexuels. Contrairement au projet de loi initial, cela tend à créer deux types de bénéficiaires de l'AMP.

et ne seront donc pas pris en charge. Est-ce juste ? Il est bon de le rappeler, l'homosexualité n'est pas un choix. Aussi, comment peut-on refuser cette prise en charge solidaire par la sécurité sociale à ces femmes qui souhaitent avoir un enfant ? J'ai déposé deux amendements pour corriger cette

En effet, est-il concevable de dire à une femme qui s'est engagée avec son conjoint dans une procédure d'AMP qu'elle a le choix, en cas de décès de celui-ci, entre détruire leurs embryons ou les donner à un autre couple, alors même que l'AMP est ouverte aux femmes seules et que cette personne pourrait s'engager sur une AMP avec tiers donneur En revanche, je me félicite de ce que la commission spéciale ait pu donner une réponse positive à un certain nombre d'avancées. Il s'agit, tout d'abord, de la mise en place, par l'article 14, d'un régime de déclaration préalable pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines.

Enfin, je soutiens la proposition de Mme Imbert d'autoriser, à titre dérogatoire et dans le respect des principes éthiques, le développement d'embryons jusqu'au vingt et unième jour, dans le souci de permettre des avancées dans la compréhension du développement embryonnaire.

J'en viens maintenant à la médecine foetale et au diagnostic préimplantatoire, autre sujet très sensible examiné par le Comité consultatif national d'éthique. Je dois dire que l'audition de Mme Alexandra Benachi, présidente de la Fédération française des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, a été particulièrement remarquée et a suscité une certaine adhésion. Sur ce sujet, le spectre de l'eugénisme revient fréquemment, avec la crainte de la sélection des embryons. Il est, à mon sens, infime face aux encadrements posés par l'Agence de la biomédecine. Aujourd'hui, il faut avoir souffert pour bénéficier d'un diagnostic prénatal. C'est le terrible constat posé par Mme Benachi. à l'heure actuelle, le diagnostic préimplantatoire pour la recherche d'aneuploïdies (DPI-A) ne peut être réalisé que pour rechercher une pathologie génétique ciblée dont est porteur l'un des parents. Cela signifie qu'il faut d'abord avoir un enfant gravement malade pour pouvoir vérifier que les suivants ne le sont pas. L'avantage du DPI-A est multiple : il permet d'éviter de recourir à une interruption de grossesse, de ne pas stimuler plusieurs fois une patiente déjà âgée, mais également d'éviter des fausses couches ainsi que l'exposition à des risques de thrombose ou de cancer à long terme.

Je regrette cependant que, pour des conditions de recevabilité financière de l'amendement au regard de l'article 40 de la Constitution, ce DPI-A ne puisse être pris en charge par l'assurance maladie obligatoire, alors même qu'il augmente les résultats d'AMP.

Il n'est pas responsable de maintenir l'interdiction absolue des tests génétiques commerciaux, puisque cela permet aujourd'hui à des sociétés étrangères d'engranger des données génétiques personnelles en dehors de tout contrôle et sans conseil délivré par des professionnels qualifiés.

Pourtant, de vraies questions éthiques se posent avec le développement des nanoparticules, de la notion d'effet cocktail et la latence des polluants. Pour conclure, je souhaite que nous puissions débattre sereinement de ces problèmes éthiques parfois très complexes, mais qui recouvrent des réalités très concrètes pour nos concitoyens. nos concitoyens. Montesquieu a écrit : « Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie ; il ne faut pas être au-dessus des hommes, il faut être avec eux. » Alors, soyons curieux, écoutons-nous, respectons-nous, afin d'élaborer ensemble un texte juste, qui soit le reflet des évolutions de notre société et qui anticipe celles à venir. La

en matière de bioéthique, nous ne partons pas de rien ! C'est en effet la cinquième fois que nous légiférons, en comptant la loi de 2013 relative à la recherche sur l'embryon humain. Il y a un peu plus de vingt-cinq ans, j'ai eu le privilège d'être associé à l'élaboration des premières lois de bioéthique, aux côtés de Simone Veil. Le sujet était alors entièrement à défricher, et la France se voulait pionnière. Aujourd'hui, nous disposons d'une législation de bioéthique moderne et unique au monde. Il me semble que nous ne devrions la modifier que d'une main tremblante, en sachant préserver ses principes fondateurs. En 1993, nous ignorions bien sûr quels seraient les développements à venir des sciences du vivant. Mais, justement, le Parlement a voulu poser des principes à l'épreuve des temps, des principes qui ne seraient pas subordonnés à l'état de la science. Ces principes expriment d'abord une vision de l'homme et des valeurs de notre société. Ils ne sont pas contingents. Ils se veulent au contraire permanents, et même intangibles : primauté de la personne humaine respect de la dignité de l'être humain dès le commencement de la vie ; interdiction de toute discrimination fondée sur des caractéristiques génétiques ; interdiction de la création d'embryons humains pour la recherche et encadrement strict de celle-ci intégrité de l'espèce humaine et, donc, interdiction de toute pratique eugénique reposant sur la sélection des embryons humains refus de toute manipulation du génome humain, ce qui implique bien sûr l'interdiction de la création de chimères, c'est-à-dire de cellules hybrides, en partie humaines, en partie animales ; enfin, indisponibilité du corps humain et de ses éléments, parce que le corps n'est pas une chose, il est la personne même et l'homme ne peut pas en faire ce qu'il veut. C'est aussi ce qui rend incompatibles avec notre civilisation l'esclavage, le contrat de prostitution ou la gestation pour autrui. Ce sont des règles fondamentales. De l'aveu même du Conseil constitutionnel, elles concourent au « respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine », ce qui n'est pas tout à fait secondaire en matière de droits fondamentaux Cela n'interdit pas de faire évoluer les modalités d'application de ces principes. Mais, pour l'essentiel, notre devoir me paraît être de les conforter et non de les fragiliser. L'idée qu'il faudrait changer nos principes en fonction des besoins de la recherche porte en elle la négation même de ces principes, un peu comme si nous devions réviser régulièrement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour l'adapter à de nouvelles exigences. Ce serait une façon de s'en remettre par avance au principe d'utilité, admettre que désormais utilité fait loi. Est-ce bien la société que nous voulons ? En matière d'éthique des sciences du vivant, le choix français est de confier au législateur le soin de décider lui-même ce qui est permis et ce qui est interdit. Ce n'est ni aux savants ni aux médecins de le faire. Ils seraient en outre juges et parties. C'est au Parlement que revient la responsabilité, et c'est une bien lourde responsabilité. Je suis heureux que notre commission spéciale, après s'être donné le temps de la réflexion, ait opté aujourd'hui pour une certaine prudence face aux tentations prométhéennes en matière de recherches et aux risques de dérives eugéniques. Des recherches strictement encadrées sur des embryons humains surnuméraires qui ne font plus l'objet d'un projet de grossesse sont déjà autorisées dans des limites qui ont été assouplies par les lois de bioéthique et par la loi de 2013. Toute demande d'un nouvel élargissement ne peut être examinée qu'avec la plus grande circonspection. Les cultures de cellules embryonnaires humaines ne doivent pas être banalisées, pas plus que la création de cellules pluripotentes à partir de cellules humaines adultes. Notre rôle n'est pas de nous prononcer sur la dimension scientifique de ces questions, est de fixer un cadre, des limites et des procédures apportant des garanties. La prévention des dérives eugéniques devrait également mobiliser toute notre attention. Avoir un enfant indemne d'une maladie génétique héréditaire mortelle grâce à l'identification d'un embryon non porteur de cette maladie me paraît légitime quand on a perdu un enfant d'une telle maladie ou quand on a la certitude d'un risque très élevé d'avoir un enfant atteint. Aller au-delà nous exposerait à une sélection génétique en décidant à partir de quand une vie vaut d'être vécue et pourrait conduire un jour à autoriser le choix de certaines caractéristiques de l'enfant à naître, en particulier celui du sexe. Ce n'est pas une vue de l'esprit quand on connaît les demandes qui s'expriment dans notre société et quand on observe les pratiques qui se développent ailleurs qu'en France. De la même façon, nous devons être vigilants quand il s'agit de déclencher une grossesse pour faire naître, à partir d'un tri d'embryons, un enfant susceptible d'être un donneur de sang de cordon compatible avec un frère ou une soeur atteint d'une maladie génétique grave et incurable, qu'on espère ainsi pouvoir sauver. Cette possibilité a été ouverte par la loi de 2004 et étendue en 2011. Il me semble que nous devrions nous en tenir là ! Reste la question qui mobilise l'intégralité du débat public autour de cette loi. Ce n'est pas une question de bioéthique, c'est une pure question de société. Faut-il autoriser le recours à la fécondation autrement que pour remédier à une infertilité ? En ce qui me concerne, je n'y suis pas favorable. Lors du vote des premières lois de bioéthique, le premier « bébé-éprouvette » français conçu avec donneur avait 12 ans. Nous n'avions à l'époque aucune expérience de ce que seraient l'adolescence et le passage à l'âge adulte de ces enfants. Nous en avons maintenant, et nous savons que, dans un nombre élevé de cas, alors même que tous ces enfants ont ou ont eu un père, le besoin d'un accès aux origines, que nous allons traiter dans ce texte, s'est exprimé avec force comme un cri, comme une souffrance. On peut penser qu'une faille s'est progressivement creusée dans la personnalité de ces enfants, de manière invisible aux yeux des parents eux-mêmes, une faille que l'amour et les qualités éducatives de ceux-ci n'ont pas suffi à combler. Nous devrions être humbles devant l'étendue de notre ignorance et devant notre manque de recul. Les jeunes femmes qui veulent avoir un enfant seule ou à deux par une fécondation devraient essayer d'être prudentes elles aussi, quelle que soit l'intensité de leur légitime désir d'enfant. si la recherche des origines peut revêtir une telle importance pour la construction psychique d'enfants qui ont un père, combien plus importante sera nécessairement la recherche d'un père pour des enfants auxquels on aura dès leur conception et de propos délibéré refusé d'en donner un ? Devons-nous le permettre en dépit de cette inquiétude pour le développement de l'enfant Bien sûr, on pourrait considérer que cette décision doit relever de la liberté de conscience de chaque femme. Nous pourrions à la fois exprimer de fortes objections à cette pratique et accepter de ne plus l'interdire. Ce raisonnement à l'anglo-saxonne n'est sans doute pas dénué de mérite, mais je préfère raisonner à la française, en considérant que la loi doit servir de référence aux comportements individuels et protéger l'enfant à naître.

On vient de le rappeler : depuis 1994, nous, parlementaires, sommes amenés à inscrire dans la loi la façon dont la société entend encadrer les pratiques médicales et la recherche sur la vie. L'enjeu est de taille : trouver un point d'équilibre pour mieux soigner, pour ne pas freiner les innovations scientifiques, tout en veillant à protéger le plus précieux, notre humanité. Tel est notre rôle, et il n'est pas simple. Ne perdons pas de vue que, quotidiennement, des équipes de soignantes et de soignants ainsi que des équipes de chercheurs s'attachent à prendre les meilleures décisions dans le respect des grands principes bioéthiques patient et le respect de sa décision ; ensuite, la non-malfaisance, pilier de la pratique médicale depuis Hippocrate, et son pendant, la bienfaisance, qui vise le mieux-être du patient et du plus grand nombre enfin, la justice, qui place la décision prise au regard des conséquences sur la société dans son ensemble, principe qui fait appel à la solidarité, par exemple pour la prise en charge financière et l'égalité devant l'accès aux soins.

en matière de bioéthique. L'ouverture aux couples de femmes et aux femmes seules de l'assistance médicale à la procréation va jalonner le long chemin vers l'égalité ; elle ne présente rien d'innovant sur le plan de la réflexion éthique. de grandes avancées sur le plan de l'égalité entre toutes les femmes et constitue une nouvelle étape du droit des femmes à disposer de leur corps. Au-delà, ce texte de loi se doit de répondre aux nouvelles questions éthiques. Premièrement, la recherche sur le génome et les tests génétiques ont progressé, et nécessitent d'être encadrés : le consentement à ces examens génétiques devra être recueilli et la communication de résultats ne s'effectuera que sous couvert de prévention ou de soins. Deuxièmement, dans le cas de fécondations, des diagnostics anténataux permettent aujourd'hui de détecter d'éventuelles maladies génétiques avant de procéder à l'implantation de l'embryon. Les socialistes proposeront, à titre expérimental, de diagnostiquer d'éventuelles aneuploïdies, anomalies portant sur le nombre de chromosomes, qui, pour certaines, aboutissent à des fausses couches évitables.

projet parental, il nous semble pertinent d'expérimenter cette technique, conformément aux souhaits formulés par les gynécologues auditionnés. Par ces techniques innovantes et leur pratique ainsi clairement encadrée, nous estimons pouvoir

Il n'en est absolument pas question. D'immenses précautions sont prises pour écarter les risques de discrimination, de sélection d'embryons avant la grossesse ou encore de modification génomique sans but thérapeutique. La bioéthique porte sur les sciences de la vie et de la santé. Elle nous rappelle que l'éthique s'enracine dans des activités concrètes, au fondement de la vie, de la médecine et du soin, pour sauver des vies humaines menacées et fragiles, pour lutter contre la maladie et contre la mort. Comme le dit Jacqueline Mandelbaum, ancienne membre du Comité consultatif national d'éthique, la bioéthique est là pour « réfléchir ensemble, prendre du champ, du temps, jeter le doute dans la mare de nos certitudes, ne jamais oublier l'autre, l'humain, caché derrière le mirage technologique ou la force du désir Chers collègues, dans les jours à venir, nous allons confronter nos visions, nos convictions, nos certitudes. Aiguillonnés par les attentes de nos concitoyennes et de nos concitoyens, nourris de nos doutes et de nos espoirs, nous allons ouvrir l'éventail de la pratique médicale et de la recherche biologique. Nous allons aussi fixer des limites, tracer des frontières et ainsi contribuer à définir l'espace où se loge l'humanité, dans la promesse infinie de la technologie. Soyons à la hauteur !

De ce point de vue, toute disposition visant à inciter les donneurs potentiels et à les rassurer est la bienvenue, même s'il serait nécessaire d'aller plus loin. Je vais y venir. Concernant le statut du donneur, il faut saluer l'initiative de notre commission spéciale, qui a le mérite de poser le principe. Mais des mesures complémentaires pourraient être étudiées, notamment afin de garantir le principe de neutralité financière : si le don ne peut en aucun cas rapporter au donneur, il ne doit pas pour autant lui coûter. je pense à la réduction des délais de remboursement des frais exposés par les donneurs, à leur exonération du ticket modérateur, ou encore à l'interdiction des dépassements d'honoraires pour leur prise en charge. Sur ces questions, les amendements de notre collègue Daniel Chasseing sont les bienvenus. Plus ambitieux est l'article 5, qui a vocation à lever les contraintes pesant actuellement sur la pratique du don croisé, afin de dépasser les cas d'incompatibilité biologique entre un receveur et un proche disposé à consentir au don d'organes. Créé par la loi de 2011, le don croisé n'a été que peu mis en oeuvre, en raison notamment de la limitation du nombre de tandems de donneurs et de receveurs mobilisables, et sans doute aussi du fait de l'exigence de simultanéité des opérations de prélèvement et de greffe, qui requiert non moins de quatre blocs opératoires. le texte de la commission rétablit opportunément à six le nombre de paires mobilisables. De même, il met fin à l'exigence de simultanéité en introduisant un délai maximum de vingt-quatre heures pour la réalisation des opérations de prélèvement et de greffe.

Les articles 6 et 7 renforcent quant à eux la protection des mineurs et majeurs protégés dans l'expression de leur consentement aux dons, précaution à laquelle on ne peut que souscrire. des États généraux de la bioéthique et l'avis du Comité consultatif national d'éthique, présentés en 2018, avaient en effet insisté sur l'attention à porter à ce consentement, notamment au regard des pressions intrafamiliales, évoquées devant nous par le grand rabbin de France, Haïm Korsia. l'article 7 étend aux mineurs de 17 ans la possibilité, en l'encadrant, de participer aux opérations de don du sang. Cette extension est logique, au regard des campagnes d'information et de sensibilisation conduites auprès des 16-18 ans dans le cadre de la journée défense et citoyenneté. Au-delà des aspects législatifs, il me semble nécessaire de maintenir et de renforcer l'information sur le don, qu'il s'agisse de son cadre juridique, de la présomption de consentement ou encore du protocole dit « Maastricht III », concernant le prélèvement d'organes dans le cadre d'un arrêt des soins. La question de l'égalité territoriale pour l'accès aux dons me semble également essentielle. Je pense notamment aux différences constatées en matière d'inscription des patients sur liste d'attente de greffe, même si une liste nationale d'urgence Enfin, les problématiques des greffes pratiquées à l'étranger et du trafic d'organes doivent trouver une solution. Les élus de notre groupe proposeront des amendements en ce sens : j'espère que ces dispositions seront adoptées, tant ces pratiques comportent de risques, pour les donneurs comme pour les receveurs.

prétention scientifique et encore moins moraliste ; mais, en tant que parlementaire et comme citoyenne, je vous livrerai certaines interrogations, qui, parfois, soulèvent des inquiétudes.

portée. Permettre à toutes les femmes de mener à bien leur projet familial en toute légalité est une avancée pour notre pays. Cette mesure aurait pu être examinée dans un autre projet de loi, plus sociétal ... C'est vrai ! En effet, son caractère bioéthique apparaît quelque peu discutable. Quoi qu'il en soit, demain, avec l'adoption de ce texte, notre législation dira : le cadre familial peut être multiple et nous reconnaissons l'entité familiale dans cette multiplicité, le mythe de la famille idéale ne résistant d'ailleurs à aucune étude. C'est en prenant acte de cette même réalité que le droit à la filiation évolue aujourd'hui, même si, selon nous, la reconnaissance conjointe anticipée devrait être étendue à tous les couples ayant recours à l'AMP, et non seulement seulement aux couples de même sexe. Les deux régimes différents que défend le Gouvernement ne se justifient pas. Nous proposerons des amendements en conséquence. Le texte issu de la commission spéciale est globalement satisfaisant en matière de procréation ; mais d'autres avancées importantes sont aussi à souligner. Dans le cadre du triptyque constitué par les principes de dignité, de liberté et de solidarité, un encadrement éthique a été fixé pour plusieurs évolutions techniques et technologiques. Je pense à l'intelligence artificielle, avec la consécration du principe d'une garantie humaine dans l'interprétation des résultats en cas d'utilisation d'un algorithme et l'encadrement du recours à l'enregistrement de l'activité cérébrale. Je pense également au renforcement du consentement et de l'information concernant les découvertes

que tout don provenant du corps humain- organes, cellules, tissus -s'effectue en toute gratuité. De surcroît, le don croisé d'organes

Au lieu de multiplier les précautions, ne serait-il pas plus judicieux de réfléchir aux moyens que nous devrions déployer pour la mise en oeuvre d'une véritable politique familiale ?

Dans un monde toujours plus pollué, dans lequel nous travaillerons, demain, de plus en plus longtemps- c'est en tout cas ce qu'envisage le Gouvernement avec la réforme des retraites -, l'on nous propose de repousser nos limites naturelles en conservant l'option, surtout pour les femmes, de faire un bébé « en temps et en heure », ou plutôt dans une fenêtre spatio-temporelle qui relèvera non plus de la biologie humaine, mais des impératifs sociétaux et libéraux. Ma réflexion va un peu loin, mais il me semble nécessaire de la pousser ainsi,

Encore interdite en 1994, en vertu des premières lois de bioéthique, la recherche sur embryons humains est aujourd'hui proposée dans un cadre très large. Elle répond non plus forcément à des buts médicaux, mais à un souci de connaissance biologique.

En encadrant les expérimentations impliquant la création d'embryons chimériques par l'adjonction de cellules souches pluripotentes humaines à un embryon animal, la commission spéciale du Sénat autorise, de fait, la pratique. Or l'inquiétude est forte quant au risque de franchissement de la barrière des espèces. Ce sujet, quelles qu'en soient les possibilités offertes pour la recherche, est lourd de conséquences. Il mériterait une réflexion bien plus poussée, dans un cadre international, et pourquoi pas sur l'initiative de notre pays. Voilà ! Mes chers collègues, à l'évidence, ce qui est techniquement possible n'est pas toujours éthiquement souhaitable : c'est déjà ce que relevait Jean-Jacques Rousseau au siècle des Lumières dans son. Très bien ! Toutes les Toutes les interrogations que Rousseau soulevait alors peuvent aujourd'hui être transposées dans un double questionnement sur le progrès scientifique et l'émancipation humaine. Aujourd'hui, le débat ne peut être ni binaire ni clivant.

sûr, nos lois de bioéthique doivent évoluer, car notre société évolue ; mais selon nous, il faudrait presque les remanier comme l'on touche à la Constitution, d'une main tremblante, avec prudence et avec sagesse

les questions éthiques renvoient à la réflexion politique de chacun d'entre nous de la manière la plus intime. Elles sont alimentées par des convictions philosophiques ou encore spirituelles. Elles interrogent notre relation à l'être et le prix que nous attachons à la vie humaine. Les sénatrices et sénateurs du groupe Union Centriste se sont particulièrement impliqués, depuis plusieurs mois, dans la perspective de l'arrivée de ce texte au Sénat, et ils exprimeront leur diversité dans le débat comme lors des votes. un point de vue notoirement différent de celui de notre collègue Élisabeth Doineau. Nous voici donc aux prémices de l'examen d'un texte qui touche à des domaines très variés. En préambule, Christiane Taubira répondant aux questions des sur France 2, en octobre 2015 à propos de l'ouverture de la PMA aux couples de femmes. « Oui, je pense qu'il serait bon que nous puissions avoir le débat. Ceci étant, depuis deux ans et demi je dis que ce n'est pas simple. Ce n'est pas du " oui " ou du " non ", ce n'est pas du " pour " ou du " contre ". C'est un sujet médical, c'est un sujet important, c'est un sujet qui a des effets également sur la sécurité sociale, donc il faut le traiter en tant que tel.

Je regrette donc vivement que des mesures concernant l'établissement de la filiation, lesquelles relèvent du droit civil et ne sont pas, à proprement parler, de nature bioéthique, soient celles qui vont nous occuper le plus longtemps dans les débats et qui auront le plus grand écho médiatique.

Le droit doit, autant que faire se peut, correspondre à la réalité. Il ne doit pas constituer une fiction. C'est pour moi un élément extrêmement important, en particulier pour le recours à l'assistance médicale à la procréation. En effet, à l'absence de père, on ajoute un mensonge, une tromperie, de surcroît protégée par la loi.

je suis catégoriquement opposé à la gestation pour autrui. Je pense même que notre pays s'honorerait de prendre la tête d'une interdiction internationale, tant les exemples, notamment en Asie, démontrent que la marchandisation industrielle du corps humain peut conduire à une véritable abomination. Au moment où le cerveau est, en termes médicaux, un continent encore très largement inexploré, au moment où nous savons que des échanges très forts se produisent entre un enfant et sa mère au cours de la vie intra-utérine, je vous assure que les arguments ne manquent pas.

sa décision élude la responsabilité des parents qui y ont eu recours. Ce sont eux qui mettent leurs enfants dans une telle situation : la faute ne peut incomber au législateur français, qu'il est tellement facile d'incriminer Aujourd'hui, on évoque des verrous : j'ai bien peur que ces verrous ne deviennent demain des cliquets et qu'ils ne nous conduisent progressivement vers la légalisation de la GPA dans notre pays. L'application dévoyée du principe d'égalité nous conduira là, et les fondations seront déjà bien installées dans notre droit.

Le législateur, s'il représente le peuple, ne doit jamais céder à l'opinion publique, d'autant qu'elle est très évolutive : ce qui est acceptable aujourd'hui peut ne plus l'être demain.

n'en va pas moins, à bien des égards, plus loin que celui de l'Assemblée nationale, et fait sauter au passage des garanties posées par les députés. Qu'il s'agisse de la question des chimères, du régime juridique des embryons ou des cellules souches, des bébés-médicaments ou du diagnostic préimplantatoire, les sujets de préoccupation ne manquent pas. La préservation de la dignité humaine doit être notre seule boussole. suppose parfois de fixer des limites en s'engageant à ne jamais les franchir, quand bien même la recherche médicale le proposerait. C'est tout l'enjeu de ce texte ; c'est la raison pour laquelle les membres de mon groupe prendront part aux débats avec la liberté et la responsabilité personnelles qui les caractérisent. De tous ces sujets, nous reparlerons

monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, pour ce texte relatif à la bioéthique, dont nous engageons aujourd'hui l'examen, nous avons toutes et tous reçu de très nombreux courriers de particuliers, d'associations et de professionnels, tant en accord qu'en désaccord, et ce de façon transpartisane. Il n'aura échappé à personne que ce projet de loi suscite beaucoup de polémiques. Pour tenter d'y répondre, la commission spéciale chargée d'examiner ce texte a auditionné, de façon très large, des représentants de courants de pensée,

aujourd'hui, en 2020. Je pense non seulement aux différentes positions concernant l'AMP, sujet d'ailleurs plutôt de société que de bioéthique, ... C'est vrai ! ... mais aussi aux progrès de la recherche, attendus pour beaucoup. Cette tâche fut d'autant plus délicate que les vifs désaccords des années 1990 perdurent.

ni le fait que les actes mentionnent la mère ayant accouché et une autre femme ne font obstacle à leur transcription, dès lors que ces actes sont réguliers dans le pays dans lequel ils ont été établis. Comment ne pas légiférer dans ce sens par la suite ? Nous pouvons difficilement aller à l'encontre du fait que toute femme a la capacité de porter un enfant et de le désirer. Nous ne pouvons plus laisser des femmes qui le désirent ardemment aller à l'étranger pour bénéficier d'une aide médicale à la procréation. Certains diront que, avec la légalisation de l'AMP pour des schémas familiaux différant de ceux que nos parents ont pu connaître, nous faisons le deuil de la famille traditionnelle. Mais combien de familles sont déjà monoparentales ? Dans le département dont je Dans la plupart des cas, l'enfant vit alors entre deux parents, qui ne forment en aucun cas une unité parentale. L'important n'est-il pas un environnement aimant et solide, qui permette à l'enfant de s'épanouir ? Mais, bien entendu, autoriser l'AMP n'est pas autoriser la GPA : les deux ne peuvent être assimilées ! Nous devons nous attacher à déployer tous les garde-fous afin d'empêcher les dérives. C'est ce que la commission spéciale s'est employée à faire, sur la proposition de ses rapporteurs : elle a affirmé l'interdiction de la gestation pour autrui en France. Elle a également rappelé la nécessaire notion d'infertilité pour l'accès à l'AMP des couples hétérosexuels et interdit le double don de gamètes. concernant l'accès à l'identité du donneur, elle a été soucieuse du respect de la vie privée, en demandant un accord exprès du donneur au moment de la demande du receveur devenu majeur. Toutes ces mesures me semblent bien encadrer l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules, tout en comblant des failles existantes dans la procédure déjà en place de l'AMP pour les couples hétérosexuels. Pour reprendre les termes d'un pédopsychiatre que nous avons auditionné, ce sont là autant d'enfants « à qui nous ne mentirons plus ». Au sujet de la filiation, je soutiendrai l'amendement de ma collègue Sophie Primas. Il vise à préserver la filiation actuelle

Elle s'est attachée à la gratuité du don, a créé un statut du donneur d'organe et permis le don de son sang dès l'âge de 17 ans. Ces apports me semblent très intéressants.

souhaitée par le Sénat, permet de nombreux ajustements pour que soient en harmonie les évolutions parallèles de la science, d'une part, et les besoins de notre société, d'autre part.

Si l'histoire est un processus de changement lent et profond des organisations sociales et des consciences, chacun sait qu'elle est constituée de points de bascule, de changements de configuration sociale. Monsieur le président Retailleau, c'est ce que vous

depuis 1966. Le recours au tiers donneur pour la procréation ne date pas d'hier : depuis 1973, des dizaines de milliers d'enfants sont nés ainsi, au rythme d'environ mille par an. Ce progrès de l'AMP a été encadré par un corpus législatif dont le modèle est toujours calqué sur la procréation naturelle et qui rend le don invisible, au profit d'une fiction organisée par la loi. Il faut faire comme si le père était le géniteur, au prix d'un secret de famille délibéré. Combien, dans cet hémicycle, ont eu recours à ce procédé ? Combien l'ont assumé devant leurs enfants ?

Pourquoi leur refuser la prise en charge par la sécurité sociale ? Pourquoi soutenir cette inégalité de fait entre deux parties du genre humain ?

collègues, au sein de la commission spéciale, les débats ont été nourris, de grande qualité et respectueux des points de vue des uns et des autres. Je ne m'en suis pas caché, je suis contre l'extension de l'accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Pour autant, je suis favorable à plusieurs dispositions contenues dans les titres II, III et IV, relatives à la diffusion de nouveaux progrès scientifiques et technologiques et en lien avec la médecine génomique.

des articles relevant davantage de questions sociétales et d'autres fixant de nouvelles règles pour tenir compte des avancées scientifiques. Si ce projet de loi est adopté,

Je partage maintes observations formulées par Mme Muriel Jourda, et je voudrais ici m'attarder sur le titre I et sur les conséquences, du point de vue de l'enfant, de l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules.

Rien n'est dit quant à l'intérêt de l'enfant d'être privé de père. Le droit de l'enfant à avoir un père, posé par l'article 7 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, est remplacé par le simple droit de connaître son donneur. Or, si l'on peut comprendre le désir de maternité chez toute femme, quelle que soit sa situation, il faut aussi tenir compte du droit de l'enfant à avoir un père et une mère, dans la mesure du possible.

ne trouvent pas de raison particulière de s'opposer aux nouvelles formes de parentalité, et les études scientifiques nationales et internationales ne semblent pas, à ce jour, rapporter de différences significatives et d'impact avéré sur le devenir de l'enfant. ces données ne sont guère convaincantes sur le plan méthodologique, en termes de nombre de cas et de durée d'observation d'enfants n'ayant pas toujours atteint l'âge des questions existentielles. Mes chers collègues, tout le monde s'accorde à reconnaître que les rôles des mères et des pères ne sont pas équivalents et qu'ils participent tous deux à la construction de l'identité de l'enfant. Dans le cas d'une AMP pour un couple de femmes,

L'enjeu, pour l'enfant issu d'une AMP, est donc l'élaboration imaginaire de la figure paternelle, nécessaire à sa construction identitaire. En permettant l'accès aux origines, ce projet de loi recourt à une logique du parent et du donneur. La levée de l'anonymat situe chacun à sa place et permet à chacun des contributeurs aux origines de l'enfant de jouer pleinement son rôle de support d'identification. Cependant, si ouvrir l'accès aux données non identifiantes du donneur pourrait être une mesure satisfaisante, j'observe que, dans la très grande majorité des cas, les enfants nés d'une AMP ne cherchent pas à connaître l'identité du donneur.

Sylviane Agacinski le dit très bien : tout est justifié au nom des intérêts individuels et des demandes sociétales, que le droit est sommé de ne pas entraver. Bien que le Gouvernement nous assure du contraire, je crains que l'application du raisonnement « égalitaire » dans des champs où il ne devrait pas intervenir n'amène tôt ou tard à encadrer également la demande des hommes seuls ou en couple par des techniques et des lois.

que le droit pose pour protéger l'être humain face à " l'appétit " des chercheurs. Or, le principe de la liberté des chercheurs ne porte aucun caractère absolu. Il doit être concilié avec d'autres principes, voire écarté quand est en cause la substance même du principe de dignité ». Il appartient donc à la science Il appartient donc à la science de dire ce qui est et au législateur de fixer des règles et des principes qui doivent encadrer cette recherche pour protéger les individus. Alors que le principe de précaution est consacré en matière de droit de l'environnement depuis la loi Barnier du 2 janvier 1995,

indique que « les progrès de la biologie et de la médecine doivent être utilisés pour le bénéfice des générations présentes et futures ». Consciente que les décisions portant sur les questions éthiques que posent la médecine, les sciences de la vie et les technologies associées peuvent avoir un impact sur les individus, les familles, les groupes ou communautés et sur l'humanité tout entière, l'Unesco a souhaité affirmer, dans la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme du 19 octobre 2005, que « l'incidence des sciences de la vie sur les générations futures [ ...] devrait être dûment prise en considération du principe de précaution connaît aujourd'hui un développement hors du terrain du droit de l'environnement. En France, ce principe a été introduit dans la Constitution par l'article 5 de la Charte de l'environnement de 2004. S'agissant de son champ d'application, l'article 5 vise exclusivement un dommage affectant l'environnement. Cependant, le Conseil constitutionnel pourrait tirer du texte constitutionnel la reconnaissance d'un principe général de précaution susceptible de s'appliquer dans d'autres domaines, d'autant que l'article 1 de la charte précitée lie l'environnement et la santé. Dès lors, il est tout à fait opportun de préciser dans la loi que la bioéthique est soumise au principe de précaution. La parole est

mais d'action, qui oblige « à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».

partage l'avis de Mme la rapporteure. Tout le monde admet qu'il n'y a pas de droit à l'enfant. Le Conseil d'État, dans l'avis

L'intérêt supérieur de l'enfant, c'est ce qui vient lorsque l'enfant est là, mais pas au moment de sa conception par les parents ou de l'élaboration du projet parental. Indiquer dans la loi qu'il n'y a pas de droit à l'enfant peut conduire à toute une série d'autres débats. Ainsi, lorsque dans

Il n'y a pas que les désirs des grands, il y a aussi l'intérêt de l'enfant, et cet intérêt est supérieur, dans la mesure où l'enfant est un sujet de droit vulnérable. Il semble ainsi fondamental de rappeler en préambule de ce texte que c'est l'intérêt de l'enfant qui doit primer. Trop souvent, nous faisons évoluer les lois en écoutant une partie de la population- les adultes -, sans prendre le soin d'écouter suffisamment les enfants, qui ont des droits. Ces derniers ne peuvent être assujettis au désir des parents, fussent-ils généreux.

dispose que, « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale

En réalité, le concept de primauté implique que nous prendrons toujours l'intérêt supérieur de l'enfant comme critère unique de choix, sans essayer de le mettre en balance avec d'autres. Or tel n'est pas le cas aujourd'hui

à l'enfant, mais aussi à créer délibérément des orphelins de père. Je m'oppose donc fermement à ce projet de loi, qui a pour seul objet de satisfaire à tout prix un désir d'enfant. Chers collègues, vous l'aurez compris, je suis, comme M. de Legge, contre le droit à l'enfant, mais très favorable aux droits de l'enfant. D'ailleurs, les textes internationaux invitent à protéger l'enfant et à tenir son intérêt supérieur pour une considération primordiale, comme l'a précisé M. Retailleau. La référence à l'intérêt supérieur de l'enfant dans ces traités renvoie à l'objectif de protection de l'enfant à l'échelle internationale. L'amendement de M. de Legge ayant été adopté, je retire le mien. L'amendement

les couples de femmes ne sont pas dans la même situation que les couples hétérosexuels. Ce n'est pas moi qui le dis : c'est la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Cette question de droit a été tranchée et cela figure dans l'étude d'impact du Gouvernement de façon tout à fait explicite.

à savoir l'élargissement de l'accès à la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules. Pour faire bonne mesure, les députés ont bien précisé que la PMA ne peut faire l'objet d'aucune « différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l'orientation sexuelle des personnes ». Dans sa hâte à légiférer dans le sens « progressiste », l'Assemblée nationale a laissé au Sénat le soin de de réintroduire dans le texte la situation pathologique ouvrant aujourd'hui accès à la PMA, afin que ce critère puisse continuer à s'appliquer aux couples hétérosexuels obligés d'y recourir pour cause d'infertilité. Toujours pour faire bonne mesure, l'Assemblée nationale a décidé la prise en charge de la PMA par la sécurité sociale, quels que soient les demandeurs et leurs motivations. On dérembourse l'homéopathie à cause d'un prétendu manque d'efficacité, mais on rembourse la PMA non thérapeutique, c'est-à-dire pour convenance personnelle. Il appartiendra au Sénat, sur l'initiative de la commission spéciale, d'exclure le remboursement pour les couples hétérosexuels fertiles, les couples de femmes et les femmes seules. Reste le problème de fond : soumettre l'engendrement par PMA d'un être humain à un simple projet parental est discutable ; la légalisation de la filiation volontairement sans père est invraisemblable. Dans notre société si éprise d'égalité et de justice, comment ne pas voir l'injustice infligée à des enfants qui n'auront pas de lignée paternelle ? Telle est la raison pour laquelle je voterai pour la suppression de l'article 1. a aussi le spectre de la gestation pour autrui. À chaque fois, le Gouvernement proclame haut et fort que l'« avancée sociétale » qu'il veut faire voter sera la dernière. Mais après le PACS, on a eu le mariage pour tous ... C'est ainsi que la GPA est déjà en marche. En octobre dernier, la Cour de cassation a reconnu aux partenaires d'un couple d'hommes le droit d'être tous les deux inscrits à l'état civil français comme parents d'un enfant né à l'étranger d'une gestation pour autrui. La philosophe de gauche Sylviane Agacinski a déclaré au Sénat que cet arrêt de la Cour de cassation était « le cheval de Troie des partisans de la GPA en France ». C'est pourquoi, malgré les améliorations que le Sénat apportera à ce projet de loi, je voterai contre, car il porte en germe, pour demain, la marchandisation du corps des femmes des pays pauvres, et, pour après-demain, l'eugénisme, c'est-à-dire la sélection d'enfants parfaits.

est interdite en France pour tout le monde, car les valeurs de notre modèle sont incompatibles avec cette forme de marchandisation, d'exploitation des ventres des femmes. Il n'y a pas en l'espèce de rupture d'égalité envers quiconque.

que je comprends la souffrance de certains de mes compatriotes de ne pas avoir d'enfant : en premier lieu les célibataires, puis les couples dont la stérilité n'a pu être soignée, enfin les couples composés de deux personnes du même sexe. Pour autant, vouloir soigner cette souffrance par une conception médicalement assistée qui prive délibérément de père les enfants à naître reviendrait à dénier au père tout autre rôle que celui de simple géniteur, à nier la différence et la complémentarité des sexes, ainsi que le besoin de l'enfant de savoir qu'il est né de la relation amoureuse d'un homme, son père, et d'une femme, sa mère,

cet article est le vrai marqueur d'un projet de loi qui, dans sa globalité, comporte d'autres dérives également graves pour notre société : l'ouverture d'un marché de la procréation, le dévoiement de la mission de la médecine, avec un glissement d'une médecine

Il soulève, comme tous les textes bioéthiques qui l'ont précédé, de nombreuses interrogations, car il touche à des enjeux complexes, empreints de vécus, de points de vue

leur statut matrimonial ou à leur identité de genre. Je tiens à le redire, les Françaises et les Français y sont prêts : les deux tiers de la population s'y déclarent favorables. Si je me réjouis que nous, parlementaires, puissions enfin examiner cette mesure très attendue par de nombreuses femmes et de nombreuses familles, qui permettra à la France de rejoindre les pays européens l'ayant précédée sur ce chemin - la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas -, je regrette qu'il ait fallu tant de temps pour en arriver là. Cette extension de la PMA permettra de sécuriser le parcours de toutes les femmes qui doivent actuellement se rendre à l'étranger pour y avoir recours, dans une démarche coûteuse et éprouvante et dans des conditions médicales médicales parfois loin d'être optimales. Notre devoir est d'apporter la sécurité, y compris médicale, à ces femmes et à ces familles. Il s'agit aussi et surtout surtout de sécuriser la situation de nombreux enfants, en rendant plus facile la filiation avec leur deuxième parent. Je tiens à saluer ici le courage et la détermination dont ont fait preuve preuve celles et ceux qui, par leur lutte, ont permis que nous examinions ce texte aujourd'hui. Ne nous laissons pas entraîner dans de faux débats caricaturaux. Ne nous y trompons pas : l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, c'est l'égalité effective par les droits, l'absence de hiérarchie entre les modèles familiaux, le droit des femmes à disposer librement de leur corps, le droit au meilleur choix possible, pour leur enfant et pour elles-mêmes. Ce droit doit être accessible à toutes, car un droit auquel seules quelques-unes auraient accès du fait de leurs revenus ne serait pas un droit effectif. C'est la raison pour le remboursement de la PMA par la sécurité sociale. Mes chers collègues, soyons à la hauteur de l'enjeu et des générations futures

depuis 1994 ? Le dispositif qui nous est proposé est pour l'heure imparfait ; c'est au Sénat d'y remédier.

que 65 % de nos concitoyennes et concitoyens sont favorables à l'ouverture de la PMA aux couples de même sexe. Ne l'oublions pas : la France nous écoute Vu le temps qui m'est imparti, je m'en tiendrai à l'essentiel, bien que les « bizarreries » et les incohérences ne manquent pas dans ce texte. S'il n'autorise pas encore la gestation pour autrui, ce projet de loi lui ouvre tout grand les portes, ainsi que, surtout, à la marchandisation de l'enfant. introduite par le texte, en effet, c'est l'autorisation en France de la « conception pour autrui », la CPA, autrement dit de la fabrication d'un enfant à partir de gamètes n'appartenant à aucun de ses parents légaux autre chose, donc, que l'« assistance à la procréation » de l'actuel code de la santé publique, la PMA. Il est donc faux d'affirmer que l'on se contente « d'élargir l'accès aux techniques disponibles sans s'affranchir de nos principes éthiques ». On s'en affranchit, en effet,

des membres du couple ». L'embryon se trouve ainsi transformé en produit, et donc, potentiellement, en marchandise lestée d'un prix et inévitablement objet d'une sélection. Certes, les gamètes nécessaires à la fabrication de l'embryon et l'embryon lui-même sont censés ne provenir que de dons- parfaitement illusoire, comme le montre l'explosion de la bio-industrie partout dans le monde. Qui, en effet, faute d'offre suffisante, empêchera le trafic de gamètes et d'embryons et les gratifications, officielles ou occultes, des opérateurs, dont il faudra bien rétribuer les services et les choix ayant présidé à l'« appariement » entre donneurs et receveurs ? Qui sait d'ailleurs jusqu'où ira cette obsession de la ressemblance et quels chemins elle prendra ? La logique du broyeur libéral étant de transformer en marchandise, outre les produits de l'activité des hommes, leur travail, l'environnement et le vivant, autoriser la création puis la transplantation d'embryons sans lien autre que fantasmé avec les receveurs, c'est ouvrir tout grand la porte à la marchandisation de l'enfant. Préférant le rôle de « conservateur humaniste » prudent à celui de « progressiste mercantiliste », je ne voterai pas un texte dont personne aujourd'hui ne peut mesurer les conséquences. Je laisse à d'autres la responsabilité de ce progrès ! La

On dit souvent que les questions de bioéthique relèvent des convictions personnelles. Je ne suis pas tout à fait d'accord, dans la mesure où notre rôle, en tant que législateur, est de dénoncer toutes les menaces qui pèsent dès aujourd'hui sur les êtres humains et qui pèseront demain sur les générations futures.

et nous ne saurions légiférer trop vite, sans visibilité, sans appréhension réelle des conséquences des bouleversements que ce texte vise à engager. Nous allons modifier en profondeur la filiation et supprimer le père du modèle légal de filiation. Du point de vue des enfants, cela signifie que nous institutionnalisons, par la loi, l'absence de père. En outre, la PMA ne nous mènera-t-elle pas inévitablement à la GPA, la marchandisation du corps humain, au nom du principe d'égalité ?

Telles sont les questions que soulève ce projet de loi relatif à la bioéthique, à commencer par son volet concernant l'ouverture de l'aide médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules. Aujourd'hui, l'AMP est réservée aux seuls couples hétérosexuels, mariés ou non, souffrant d'infertilité pathologique ou présentant un risque de transmission d'une maladie génétique grave ; 24 000 enfants naissent ainsi chaque année. Avec ce projet de loi, la demande d'AMP s'inscrit dans une revendication de liberté et d'égalité dans l'accès aux techniques pour répondre à un désir d'enfant. Elle fait émerger d'autres questions, telles que celles des conséquences d'une ouverture du dispositif sur la relation des enfants à leurs origines ou de la rareté actuelle des dons de gamètes. entre 2 000 et 4 000 femmes ont recours à l'AMP à l'étranger. Nous ne sommes donc pas devant un changement de civilisation ; ces familles existent déjà. Comme souvent, la pratique a devancé le droit et les représentations symboliques.

C'est, d'abord, faire peu de cas des familles monoparentales, qui représentent un quart des familles françaises. Le modèle classique des parents mariés qui élèvent les enfants qu'ils ont eus ensemble n'est plus majoritaire en France, soulignait l'Insee dans une étude publiée mardi dernier. C'est, ensuite, un préjugé. La filiation est un fait social et culturel, et non une vérité biologique. C'est cette vérité sociale qui fonde l'humanité, avec ses réussites, ses failles, ses faiblesses. Je ne crois pas en une éthique de la nature identifiant la morale au naturel. Nous pouvons fonder la filiation sur une base plus solide que la seule procréation procréer est un acte biologique ; être parent est un acte social, affectif, institutionnel. Ainsi, l'ouverture du droit à l'AMP mettrait fin à une forme de discrimination : toute

d'une sorte de grand marché de la procréation, où l'on serait libre de programmer une grossesse, avec ou sans père, à n'importe quel moment, de congeler ses gamètes, éventuellement sous la pression d'un employeur ... Quant à instaurer l'égalité

En attendant le meilleur des mondes, pour citer Philippe Sollers, je dirai que tout est pour le mieux dans le pire des mondes possibles

Le désir d'enfant ne leur est pas venu tout de suite ; comme pour tous les parents, il a fait l'objet de discussions, d'interrogations. C'est un projet qu'elles ont construit peu à peu, en dépassant leurs peurs, leur crainte du regard des autres, des jugements de valeur et des critiques, les préjugés étant nombreux dans une société qui prône la famille parfaite et la normalité. Or qu'est-ce que la normalité, mes chers collègues ? Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé, disait Einstein ; cette phrase m'a beaucoup inspiré dans ma réflexion sur cet article. Fanny et Aurélie ont longuement hésité ... Que faire ? Comment répondre à ce désir d'enfant ? Aller en Espagne, en Belgique ? Demander à l'un de leurs amis ? Acheter des gamètes sur internet ? Quand l'enfant vient, la joie arrive et nous éclaire », écrivait Victor Hugo. Ce désir d'enfant est un droit fondamental. Il ne doit pas être confondu avec la revendication d'un droit à l'enfant.

Ainsi, c'est non pas le droit à l'enfant, mais le désir d'enfant, que le législateur peut aider à satisfaire. C'est cette question qui nous est posée aujourd'hui. D'autres invoquent l'intérêt supérieur de l'enfant. Selon la formule, devenue célèbre, du doyen Carbonnier,

Qui serions-nous si nous devions porter des jugements de valeur à l'encontre de telle ou telle famille, sous prétexte qu'elle n'entre pas dans notre vision de la « normalité » ? La pluralité des situations familiales est une réalité que nous devons considérer et accepter, sous peine de stigmatiser certains modes de conception de l'enfant.

le rattachement d'un enfant à deux lignées parentales non équivalentes lui signifie sa propre inscription dans le genre humain, universellement mixte. Il lui permet d'assumer sa propre incomplétude, autrement dit sa sexuation

C'est pourquoi je suis prudente : le vivant est chatoyant de complexité, fort et fragile à la fois. Je n'ai que des doutes ; aussi m'abstiendrai-je sur cet article. Très bien

ce droit prend sa source dans un désir tout à fait naturel, celui de transmettre de l'amour à un enfant. Dans une société où les individus sont de plus en plus autonomes et capables d'exercer leur libre arbitre, ce désir d'enfant peut devenir un absolu. À cela s'oppose le fait que nous formons une communauté. Faire communauté, qu'elle soit nationale ou simplement de vie, nous oblige à dépasser nos individualités, parfois nos égoïsmes, à renoncer à certains de nos désirs pour cimenter le collectif. Albert Jacquard le disait La liberté n'est pas la possibilité de réaliser tous ses caprices ; elle est la possibilité de participer à la définition des contraintes qui s'imposeront à tous. crains, pour ma part, que l'extension de la PMA ne crée chez les enfants qui en seraient issus des vulnérabilités, des fragilités

par exemple, permettent la GPA, mais pas la PMA. La Grèce, la Hongrie, l'Estonie sont des pays qui autorisent la GPA, mais pas la PMA pour les couples de femmes.

de la presse, on a opposé la GPA et la PMA. On a présenté la GPA comme un cheval de Troie. En tant que médecin et que parlementaire, je ne céderai pas à ce chantage de la GPA et je voterai cet article 1, qui sera amendé par la sagesse des sénateurs.

l'AMP, l'assistance médicale à la procréation, est une technique légale en France, réservée aux couples hétérosexuels.

Si nous sommes d'accord pour reconnaître que cette technique est légale, qu'elle ne nous pose aucun problème moral, qu'elle ne concerne pas le droit à l'enfant dès lors que les parents sont hétérosexuels- elle ne commence à le concerner que si les mères sont lesbiennes ou seules si l'on accepte cette technique, si l'on n'a pas de prévention contre des couples de femmes ou les femmes seules, si l'on ne pense pas que la vulnérabilité d'un enfant serait le produit de l'absence de père, comme quelques interventions le suggèrent, La vulnérabilité d'un enfant, c'est l'absence de cadre, l'absence d'amour, l'absence d'éducation et le délaissement ! Croyez-moi un père ne suffit pas à faire un cadre pour un enfant.

on ne peut pas dire que les pères ont été extrêmement impliqués dans l'éducation des enfants. Cela ne nous empêche pas d'être construits, cadrés et structurés ! Au bout du compte, ce que vous ne supportez pas, c'est l'idée que des femmes puissent élever des enfants

Les drames de la vie, les drames vécus par des couples en guerre peuvent malheureusement priver un enfant de son père ou de sa mère.

Toutefois, pourquoi aujourd'hui organiser et financer délibérément la fabrication d'orphelins de père ?

Les études dont nous disposons ne sont pas en mesure de nous démontrer la neutralité dans l'équilibre de l'enfant quand il grandit normalement entre un père et une mère.

de glissement, comme je l'ai précisé, vers la GPA, qu'on le veuille ou non. Ce qui me gêne le plus, compte tenu du manque de gamètes, c'est le risque, selon moi inéluctable, de marchandisation. C'est la raison pour laquelle, sans détailler davantage ma position, j'ai déposé cet amendement.

Aujourd'hui, l'AMP compense une infertilité. Demain, on voudrait qu'elle compense une impossibilité. Nous sommes face à un vrai débat fondamental entre deux conceptions de la vie. La première pense que les désirs individuels doivent être satisfaits à tout prix et sans aucune limite, y compris en instituant un « droit à l'enfant ». La seconde, partagée sans doute par une majorité de Français, estime que les désirs individuels doivent être soumis à certaines limites, notamment éthiques ou biologiques, et qu'il n'existe pas de droit à l'enfant, mais bien un droit de l'enfant. De plus, cet article n'est pas, contrairement aux apparences, facteur d'égalité, et ce pour deux raisons. La première est que l'assistance à la procréation est aujourd'hui une réponse médicale à un problème médical. À l'heure actuelle, l'AMP soigne une infertilité du couple hétérosexuel. Or, de toute évidence, ce ne sont pas des raisons médicales, ni même des problèmes de fertilité, qui empêchent les femmes seules ou les couples de femmes de procréer. Il s'agit tout simplement d'une impossibilité. Parler d'« égalité » ou d'« inégalité » dans ce domaine n'a donc aucun sens. La seconde raison est que les hommes, qu'ils soient seuls ou en couple, seraient de fait privés du même droit,

l'on supprime les conditions actuelles d'accès à l'AMP, qui visent des couples composés d'un homme et d'une femme vivants confrontés à une infertilité médicalement constatée ou au risque de transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une

n° 49. Ce qui est techniquement possible n'est pas forcément souhaitable. Transformer, fût-ce potentiellement, l'enfant en produit marchand pas plus qu'épuiser la Terre ne sont des progrès au sens où l'entendaient les Lumières et où l'entend encore aujourd'hui le sens commun ! Erreur, m'objectera-t-on : ce nouveau droit à l'enfant est gratuit, puisqu'il est fondé sur le don de gamètes ou d'embryons. Sauf qu'une telle mutation ne sera gratuite ni pour la société- au moment même où la prédication officielle est à la réduction des dépenses sociales, voir l'état pitoyable du système hospitalier -, ni finalement pour les bénéficiaires. Elle sera en revanche lucrative pour les praticiens, pour la technostructure du back-office, pour les détenteurs de brevets et, plus encore, pour les investisseurs, qui voient là un nouveau champ fertile de profits.

des cellules souches, des tissus et des organes à l'échelle internationale, mais elle camoufle, selon cet auteur, « les processus de commercialisation des cellules reproductives sur lesquelles s'appuie l'industrie de la reproduction assistée Pour elle, c'est la procréation assistée qui incarne le mieux ce processus de biomécanisation du vivant, « dans la mesure où il ne s'agit pas d'une médecine curative, mais bien d'une médecine méliorative, qui a pour but de dépasser les limites des corps infertiles ». En d'autres temps, on s'étonnerait que, au nom du progrès et des droits- ici, le droit inavoué à l'enfant, reconnaissons-le de la liberté et de l'égalité, une telle fuite vers l'inconnu mercantile reçoive le soutien de l'ensemble de l'échiquier politique ! J'ai bien conscience que cet amendement a peu de chance d'être voté, même par les adversaires brevetés du néolibéralisme- comprenne qui pourra !

cet article rompt l'équilibre trouvé depuis les lois de la bioéthique en 1994 entre les nécessités du progrès scientifique et la préservation des valeurs humaines et sociales fondamentales. Cette recherche d'équilibre repose sur l'idée que tout ce qui est techniquement possible n'est pas toujours socialement souhaitable, comme cela a été souligné. Deuxièmement, s'il convient de reconnaître que la notion d'égalité, dont on a beaucoup parlé, peut se trouver au fondement de cette disposition, en donnant la possibilité à tous les couples hétérosexuels comme homosexuels de satisfaire un désir d'enfant, ce principe d'égalité se heurte à plusieurs limites. En effet, si l'on permet aux femmes homosexuelles de recourir à la médecine pour procréer sur le fondement de l'égalité, il paraît nécessaire d'en faire autant pour les hommes. On ne peut utiliser le critère d'égalité pour justifier la PMA et le nier pour la GPA. De cette question en naît alors une autre : celle de la gestation pour autrui, interdite en France au nom de l'indisponibilité du corps humain. Troisièmement, l'ouverture de la PMA aux couples de femmes remet en question tout notre droit de la filiation, en le détachant

reviendrait à priver l'enfant d'une partie de ses origines biologiques, rompant ainsi l'égalité entre les enfants, dont certains seront privés de fait et en droit de leur ascendance personnelle. La parole

Aujourd'hui, l'humilité, n'est-ce pas d'accepter une grande part des règles morales, sociales, religieuses que l'humanité avant nous et pendant des siècles a reconnues pour nécessaire ? L'évidence n'est-elle pas, mes chers collègues, de reconnaître qu'il y a une loi naturelle et que celle-ci doit fonder une partie de notre droit positif ? Cette loi naturelle, sans être triviale,

Lorsque nos collègues sur toutes les travées craignent une dérive vers la GPA, ce n'est pas une fiction, c'est évidemment le chemin que nous allons suivre, du fait de la jurisprudence européenne

Où est le bien commun ? Notre rôle de législateur n'est-il pas d'essayer de déterminer ce bien commun, qui permet de faire progresser la société, de fixer des repères et de sortir de ce triptyque infini, de cette logique des désirs : « je veux, je peux, j'y ai droit » Est-ce bien notre rôle que d'étendre infiniment les droits des individus ? Il y a un droit ci, c'est le droit de l'enfant

Le droit positif, notamment issu de la loi Taubira, répond à une grande partie des sollicitations émanant du corps social. Si des évolutions sont envisagées, il s'agit de les renvoyer à un texte, qui pourrait permettre un débat parlementaire clair, portant sur toutes les modifications des modalités de l'établissement de la filiation et sur toutes leurs conséquences. Quel

les dérives vers un droit à l'enfant- je me permettrai d'y revenir -, en dépit de l'adoption de l'amendement précédent, un détournement de la médecine ou encore un glissement vers la gestation pour autrui. Tout d'abord, je veux réaffirmer ici haut et fort que l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation sera sans incidence sur l'interdiction de la gestation pour autrui, qui est antinomique des grands principes bioéthiques auxquels nous sommes tous attachés.

Sa finalité, sa conséquence peut être d'apporter davantage d'égalité, mais ce n'est pas une loi d'égalité ou de lutte contre les discriminations. Une loi de bioéthique vise vous le savez, à scruter les techniques médicales, pour les examiner au prisme de nos principes éthiques. Or la gestation pour autrui met immédiatement en tension des principes fondamentaux de notre droit, à commencer par celui qui exclut la marchandisation du corps humain. Il n'y aura donc pas, je le redis, je l'affirme politiquement et juridiquement, de glissement vers la gestation pour autrui.

a pas aujourd'hui de droit à l'enfant. Actuellement, les couples hétérosexuels qui s'engagent dans l'assistance médicale à la procréation ne disposent pas d'un droit à l'enfant. Il en est de même pour les couples, quelle que soit leur orientation sexuelle,

Il en sera de même, demain, pour les couples de femmes ou les femmes non mariées. Par ailleurs, la légitimité d'un projet mono ou homoparental a déjà été tranchée. La sénatrice Marie-Pierre de la les textes autorisent l'adoption d'un enfant par un couple marié, y compris par un couple de femmes, ainsi que par une personne seule, et ce depuis de nombreuses années. L'essentiel pour un enfant- cela a été très bien dit par Laurence Rossignol -, c'est l'affection, l'attention et le sentiment de sécurité que l'on est en mesure de lui garantir. Des recherches, des années de pratiques de nombreux pédiatres et pédopsychiatres nous apprennent que ce n'est pas tant la structure familiale qui importe, mais la dynamique familiale qui est en cours au bénéfice de l'enfant. de l'enfant. L'essentiel pour un enfant est ce besoin de sécurité, à la fois matérielle et affective. À cet égard, beaucoup d'entre vous ont parlé d'humilité. Soyons humbles, effectivement, par rapport à ces sujets

n'est pas contradictoire avec l'existence d'autres modèles familiaux, qui sont tout aussi respectables, au sein desquels un enfant peut s'épanouir. Là encore, je suis désolé de vous le dire,

Ces figures d'attachement vont bien au-delà du cercle familial restreint, voire du cercle familial tout court.

S'agissant de la question du détournement de la médecine, qu'un certain nombre d'entre vous ont évoquée, parmi lesquels le sénateur Chevrollier, il convient de rappeler que les techniques d'assistance médicale à la procréation ne soignent pas et ne guérissent pas les couples de leur infertilité : elles agissent comme des techniques de parenté, en particulier en cas de recours à un tiers donneur. Il en est de même lorsque l'indication de l'assistance médicale à la procréation est liée à l'âge de la femme, sans autre cause médicale. Dans ces deux exemples, s'il y a bien un acte médical, l'assistance apportée par le médecin est moins médicale que sociale. C'est d'ailleurs l'Académie nationale de médecine qui établit ce constat : « De la De la chirurgie plastique à la médecine sportive, nombreux sont les actes et les missions qui peuvent être confiés aux médecins, sans que la finalité soit de corriger un état pathologique ou de se substituer à une fonction défaillante ». Mesdames, messieurs les sénateurs, sénateurs, les faits sont les suivants : les grossesses résultant de procréations engagées hors du territoire national par des femmes en couple ou célibataires sont suivies en France, les enfants naissent en France et leur filiation est légalement établie en France. Aujourd'hui, le passage des frontières est réservé aux femmes les plus aisées, ce qui aboutit à une situation d'inégalité- nous aurons l'occasion d'y revenir lorsque nous débattrons de la question du remboursement de la procréation médicale assistée pour toutes les femmes.

issue d'un modèle conjugal unique. Nos citoyens y sont prêts. Le sénateur Daudigny l'a dit : ils ont même anticipé cette évolution ! Notre devoir est d'accueillir ces nouvelles formes familiales et non de les stigmatiser. Notre devoir est d'apporter de la sécurité, y compris sur un plan médical, à ces familles et à ces femmes. Notre devoir est de permettre l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées, ici, en France. Il doit s'agir d'un véritable droit réel et non d'un droit formel. Monsieur le sénateur Karoutchi, je sais que vous y êtes attaché. Pour toutes ces raisons, nous sommes défavorables, vous l'aurez compris, à ces amendements de suppression.

Merci